Je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d'un sénateur appelé à siéger au sein du conseil de surveillance et de deux sénateurs appelés à siéger au sein du comité stratégique du comité stratégique de la société du canal Seine-Nord Europe. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a proposé la candidature de M. Jérôme Bignon, pour le conseil de surveillance, et celles de M. Jacques Legendre et Mme Nelly Tocqueville, pour le comité stratégique. Ces candidatures ont été publiées et seront ratifiées, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure. heure. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour un rappel au règlement. Madame la présidente, je veux intervenir sur un problème d'actualité, lié à une loi que nous avons adoptée récemment. Voilà environ six mois, nous avons voté une réforme du mode d'élection du Président de la République, le principal

hier la première des conséquences scandaleuses de cette réforme, puisque la principale chaîne de télévision française vient de sélectionner un certain nombre de futurs candidats, laissant les autres de côté. Or, dans un régime qui prétend être véritablement démocratique, tous les candidats à une élection, surtout lorsqu'il existe une sélection par le biais des parrainages des maires, doivent être traités sur un pied d'égalité. Je proteste contre ce dévoiement de la démocratie. Certes, je suis très minoritaire dans cette assemblée, et je sais que la loi est faite par ceux qui détiennent le pouvoir.

présentée, en application de l'article 34-1 de la Constitution, par Mme Aline Archimbaud et les membres du groupe écologiste

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, si la France a quelque avance sur l'Union européenne dans la lutte contre l'exposition aux perturbateurs endocriniens, nous le devons aux chercheurs, qui ont fait valoir la notion d'« exposome

déposée par notre groupe sur l'initiative d'Aline Archimbaud est une invitation à poursuivre ces efforts, car la Commission européenne est aujourd'hui un frein, et les lobbies tentent de faire passer leurs intérêts avant la santé publique et l'environnement.

indispensable aux nouvelles règles. Nous ne pouvons en rester là ! Ces substances restent trop présentes, la question des liens entre santé et environnement est encore trop marginale dans les politiques publiques, au point que le ministère de la santé se cantonne à la gestion et aux soins, tandis que la santé environnementale a trouvé refuge au ministère de l'écologie.

progressent quatre à cinq fois plus vite que le changement démographique. Le cancer touche un homme sur deux et deux femmes sur cinq. Il aura fallu du temps pour bien identifier les mécanismes des perturbateurs endocriniens, ces petites molécules dans de nombreux produits d'usage ou de consommation courante migrent et pénètrent nos organismes, modifiant les messages normaux

si leur mère respire des solvants ou des pesticides. Il serait inimaginable de laisser sévir un mécanicien qui remplacerait les freins d'une voiture par un accélérateur

de l'appareil urogénital du foetus, imprégner les organismes, programmer des cancers du sein de la petite fille à naître, fausser la communication interne de nos organes, au risque de dysfonctionnements profonds et de maladies graves. L'vient de publier L'vient de publier une liste de 400 cosmétiques avec perturbateurs. Messieurs, votre gel douche aux parabènes et alkyphénols ne mérite pas de compromettre votre fertilité et de saboter votre descendance. Mesdames, les phtalates de votre vernis ou le benzophénone de votre teinture ne valent pas la puberté de votre fille. Bricoleurs, la rénovation de votre intérieur à grands coups de solvants ne mérite pas que vous risquiez un cancer, comme c'est le cas premières victimes des produits phytosanitaires. Après le phénoxyéthanol dans les lingettes, révélé par l'Institut national de la consommation, voici la dioxine, le glyphosate, des pesticides, des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des cancérogènes probables dans

il faut au moins un étiquetage informatif, comme nous aurions pu et dû le faire depuis un an pour les tampons et serviettes hygiéniques. Les plus jeunes sont parmi les plus exposés crèches et écoles devraient être des zones exemptes de tout perturbateur et de tout pesticide, tant dans les meubles, l'alimentation et les produits d'hygiène que dans les jouets.

ont établi les risques importants que fait peser l'usage des pesticides sur la qualité des eaux et de l'air, donc sur la santé publique. Or le bilan dressé en novembre 2015 par le Conseil général de l'environnement et du développement durable sur la qualité des eaux de notre pays fait état d'une contamination généralisée par les pesticides : dans 92 % des points de surveillance, la présence d'au moins un pesticide a été détectée et, en moyenne, 15 pesticides différents ont été recensés sur chaque point de mesure.

aux abords des zones d'habitation et des écoles. Une classe d'insecticides couramment utilisée pourrait affecter les performances cognitives d'enfants qui en ont absorbé.

Mais pense-t-on, au-delà des douleurs des personnes atteintes, aux dommages financiers ? Selon les économistes Julia Ferguson et Alistair Hunt, le coût des cinq catégories de troubles ou de maladies liés à des déséquilibres hormonaux est en France de 82 milliards d'euros annuels, sans compter les coûts induits comme l'absentéisme. Sauf à compter sur davantage de malades, donc davantage de dépenses de santé pour relancer la croissance, il faut mettre un terme à cette absurdité. Dès lors, comment agir vis-à-vis de Bruxelles ? Sans critères de définition des perturbateurs endocriniens, l'Europe ne possède pas l'outil conceptuel nécessaire pour organiser la révision de sa réglementation et agir pour la santé et la biodiversité. Elle en est réduite à des mesures de sauvegarde, qui sont certes nécessaires dans l'immédiat, mais tout à fait insuffisantes pour prendre le problème à bras-le-corps. Parce qu'elle a repoussé l'élaboration de ces critères de façon dilatoire, la Commission européenne a été condamnée le 16 décembre dernier. Sous l'influence de l'EFSA,

-et une approche fondée sur le danger, ce qui nécessite un niveau de preuve très élevé et laisse passer le risque de contaminants repérés comme probablement dangereux. Cela revient à ne pas prendre en compte le principe de précaution européen.

et de haut niveau pour une bonne instruction, par la recherche publique, du dossier européen. Il faut que les perturbateurs soient un thème de recherche prioritaire dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et le développement. si l'on doit saluer le travail associatif et ses salutaires alertes, il est paradoxal que ce dernier, qui agit à titre bénévole, informe plus vite que les instances officielles de recherche et d'évaluation. parce que les perturbateurs restent omniprésents et dangereux, parce que la France doit rester ferme, parce que ce sujet nous rassemble, je vous invite à voter cette

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de résolution présentée par notre collègue Aline Archimbaud.

cette proposition invite, souhaite, estime, considère, s'oppose, souligne. La semaine dernière, devant la commission des affaires sociales, nos collègues Patricia Schillinger et Alain Vasselle ont présenté une autre proposition de résolution, au nom de la commission des affaires européennes, sur les perturbateurs endocriniens dans les produits phytopharmaceutiques et les biocides, laquelle déplore, regrette, estime souhaite, encourage. Il s'agit, dans un cas Il s'agit, dans un cas comme dans l'autre, d'un langage propre aux résolutions. Pourtant, permettez-moi d'être un peu perplexe sur la portée de ces textes. Cherche-t-on un effet politique ou s'agit-il simplement être dans l'air du temps ? Aujourd'hui, en effet, tout le monde semble découvrir ce dossier : articles de presse et émissions télévisées se multiplient. Bref, c'est un peu l'actualité du moment. Tant mieux, dirons-nous. Voilà six ans, à la suite de l'adoption de la proposition de loi du RDSE interdisant la commercialisation des biberons produits à base de bisphénol A, j'ai réalisé un rapport sur la question des perturbateurs endocriniens. À l'époque, la terminologie elle-même était pratiquement inconnue pour nombre de nos concitoyens. Pourtant, les perturbations du système endocrinien par des substances ou des mélanges exogènes existent depuis la nuit des temps dans le milieu naturel. Certes, le développement des sciences- chimie, physique, pharmacologie, biologie -fait que, chaque jour, arrivent sur le marché de nouvelles molécules, dont les effets ne peuvent être appréciés rapidement. Pour certaines de ces nouvelles molécules, nous ne pouvons connaître d'emblée les effets nocifs dits « CMR », c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Il faut garder à l'esprit que, pour évaluer par exemple l'incidence cancérigène d'une molécule avec une certaine crédibilité scientifique, il faut une étude de cohorte, menée sur une génération. chacune de ces deux résolutions affirment, probablement à juste titre, que le principe déjà ancien selon lequel « la dose fait poison » n'est plus de mise. Pourtant, les études en laboratoire montrent des effets en courbe de Gauss pour certaines molécules, Il faut laisser du temps aux chercheurs. Selon moi, il serait parfois beaucoup plus dangereux d'interdire là où on n'a pas la certitude d'un produit de remplacement reconnu inoffensif dans la durée.

sucres, acides aminés et autres composants -, dans une approche impliquant soit un criblage ciblé large spectre des molécules, soit une recherche de molécules inattendues à partir de leur masse moléculaire. Avec l'arrivée sur le marché de spectromètres de masse à ultra-haute définition, la détection des polluants présents, par exemple dans l'eau, est faite à des doses bien inférieures au seuil réglementaire d'un microgramme par litre. Un autre point qui soulève problème est celui de la classification des substances perturbantes entre un effet néfaste supposé, suspecté ou avéré, sachant que l'évaluation évolue en permanence au cours de l'étude du produit et que les résultats ne sont pas toujours concordants selon les équipes. Je voudrais souligner l'importance de la prise en compte de la recherche scientifique mondiale sur ce dossier qui est ô combien difficile et dont l'impact économique est considérable. Depuis 1997, l'OCDE a déjà défini une dizaine de lignes directrices, afin de prendre en compte les effets mesurables des substances perturbatrices. D'autres lignes sont à définir. Elles doivent fixer un cadre permettant d'affirmer qu'une substance possède ou ne possède pas une action perturbatrice. Cela peut paraître simple, mais la réalité est tout autre selon le niveau d'informations fourni ou le niveau de complexité biologique. Des mécanismes d'action autres qu'oestrogéniques, androgéniques ou thyroïdiens sont possibles. L'effet « cocktail » est aujourd'hui avéré. Qu'en sera-t-il demain de l'action des nanoparticules et des biosimilaires ? Qu'en est-il de la valeur prédictive des méthodes de largement utilisées aujourd'hui ? Un point essentiel du débat porte sur le degré des connaissances connues sur un produit donné, le découvreur ayant théoriquement l'obligation de fournir toutes les études de toxicité conduites dans ses laboratoires. Le rôle des agences de contrôle est donc capital pour suivre ces dossiers. je le reconnais, les choses évoluent lentement et les tergiversations sont nombreuses. Quelle direction doit intervenir ? La réglementation REACH, pour, s'applique progressivement sur les substances existantes ; elle est obligatoire pour tout produit entrant sur le marché. Enfin, qu'en est-il dans notre pays ? Chacun ici connaît mon positionnement politique Je voudrais pourtant décerner un au Gouvernement, en particulier à Mme la ministre de l'environnement, pour son engagement dans la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Ce plan est bien fait : investissement dans la recherche, définition des grands axes de protection des populations les plus fragiles, renforcement de la réglementation européenne. Certes, il manque peut-être des moyens financiers suffisants. Sans doute pourrions-nous parler d'une même voix en soutenant ce plan d'action du Gouvernement. Je dois le dire, cette proposition de résolution me paraît un peu dissonante. Aussi, à titre personnel, je m'abstiendrai sur ce texte, au risque de fâcher son auteur,

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, avant toute chose, je veux remercier notre collègue Aline Archimbaud de son initiative. Mettre à l'ordre du jour de notre assemblée des sujets aussi importants que celui des perturbateurs endocriniens est utile pour la poursuite et l'enrichissement Néanmoins, ces remerciements ne s'accompagneront pas d'un soutien unanime de mon groupe à cette proposition de résolution. La santé des Français est au coeur de nos préoccupations. C'est pourquoi nous devons naturellement nous inquiéter des effets de telle ou telle substance contenue dans les produits du quotidien.

Certes, il convient d'être prudent. Toutefois, nous devons surtout faire preuve de bon sens. Le développement de produits utiles, voire nécessaires au quotidien ne peut pas se faire au détriment de la santé et de la sécurité des consommateurs ou bénéficiaires. Nous Nous ne pouvons pas faire aveuglément confiance aux industries qui développent de tels produits, c'est une évidence. Si l'immense majorité d'entre elles poursuivent leurs objectifs avec conscience et prudence, tel n'est pas le cas de quelques-unes, pour qui la recherche du profit passe avant toute autre considération. Toutefois, nous ne nous ne pouvons pas non plus tout interdire sur le simple soupçon d'un risque pour la santé ou la sécurité des consommateurs ou usagers. Sinon, plus de recherche, plus de développement, plus d'innovation ! Il ne resterait alors que la crainte de faire des erreurs, ce qu'on appelle en d'autres termes l'immobilisme. n'est pas non plus souhaitable. Aussi, que faire ? Je sais que l'on attend beaucoup des parlementaires, mais pouvons-nous réellement nous permettre d'interdire purement et simplement tel ou tel produit ? Oui, mais sous condition. Il s'agit principalement de laisser les scientifiques nous guider, en nous démontrant la dangerosité de ces produits. Si un paragraphe nous paraît très pertinent dans la proposition de résolution de notre collègue Aline Archimbaud, c'est celui qui concerne la recherche scientifique. Il faut effectivement développer la recherche sur les perturbateurs endocriniens et lui allouer des moyens financiers et humains pérennes. La coordination internationale est également essentielle à la poursuite de cet objectif. Cette recherche doit être la plus indépendante possible, car chacun ici sait à quel point l'influence de lobbies divers s'exerce par la publication de recherches scientifiques aux résultats opportunément favorables. La constitution d'un groupe international de scientifiques indépendants et de haut niveau est donc indispensable. Ce n'est qu'après la publication d'études scientifiques que le législateur peut et doit intervenir. intervenir. La commission sénatoriale des affaires européennes, dans son excellent rapport sur les perturbateurs endocriniens dans les produits phytopharmaceutiques et les biocides, n'a d'ailleurs pas manqué de le rappeler. Quant à la Commission européenne, elle a même dépassé ses compétences réglementaires en la matière, en établissant des critères de dangerosité très restrictifs et un niveau de preuve très élevé, notamment s'agissant des produits phytopharmaceutiques. Il nous paraît sage et suffisant d'appuyer les recommandations faites au Gouvernement par la commission sénatoriale des affaires européennes, à savoir le maintien d'un niveau de vigilance important dans l'élaboration de la réglementation européenne, afin d'assurer la définition de critères d'identification satisfaisants sur de nombreux produits. Mes chers collègues, nous ne voudrions pas que le trop soit l'ennemi du bien en matière de principe de précaution. Soyons donc vigilants, guidons notre action grâce au bon sens, en nous aidant des travaux menés par la recherche. Ne soyons ni hâtifs ni naïfs.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer notre collègue Aline Archimbaud, auteur de la proposition de résolution qui nous réunit aujourd'hui. Pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle ne pourra pas être présente parmi nous pour défendre son texte. Je ne puis qu'imaginer sa déception, tant elle s'est battue sur les questions de santé environnementale depuis son élection. Pour ma part, j'ai mené, depuis 2011, de nombreux combats au sein de la commission des lois pour que soient toujours protégés libertés individuelles et droits fondamentaux. Ce qui nous réunit aujourd'hui n'est finalement pas si différent. Il s'agit de permettre à nos concitoyens d'être dûment informés des substances auxquelles auxquelles ils sont exposés et de protéger la santé de toutes et tous, notamment des plus fragiles et des plus vulnérables. Cela a été rappelé, en particulier dans l'exposé des motifs de la proposition de résolution, les perturbateurs endocriniens sont, selon la définition de l'Académie de médecine, des substances ou des mélanges qui modifient le fonctionnement du système endocrinien et provoquent des effets sanitaires nocifs dans un organisme intact et sa descendance. Ils sont suspectés de provoquer des cancers hormono-dépendants, d'être reprotoxiques, d'avoir des effets néfastes sur la thyroïde, sur le développement neurologique, sur le métabolisme et sur le système cardiovasculaire. À la lecture de cette liste, on ne peut que percevoir l'immense enjeu de santé publique que constituent les perturbateurs endocriniens.

trop peu a été fait pour agir vraiment contre ce qui pourrait devenir l'une des plus grandes crises sanitaires de notre époque. Bien sûr, l'inlassable action des industriels, notamment au niveau européen, est à combattre avec la plus grande énergie. Toutefois, d'autres perspectives concrètes peuvent, et doivent, être le plus rapidement possible, tracées. Il est ainsi indispensable que la recherche universitaire sur les effets sanitaires des perturbateurs endocriniens soit plus amplement développée. Il faudrait, dès le doctorat, allouer d'importants moyens financiers et humains à la recherche publique, afin de lutter contre la désinformation propagée par les « marchands de doute que les décisions en matière de politique de santé publique puissent être prises en toute indépendance. Il est également capital que les mécanismes de contrôle de la réglementation en vigueur soient efficaces ; pour ce faire, des moyens considérables sont derechef nécessaires. En effet, aussi insuffisante que soit la réglementation en la matière, il est indispensable qu'elle soit appliquée dans les faits.

De tels investissements sont indispensables pour l'avenir. Rappelons-le : les femmes enceintes et les jeunes enfants sont les premières victimes des perturbateurs endocriniens. À ce titre, les propositions formulées par le Réseau environnement santé en vue de l'élection présidentielle sont tout à fait intéressantes. Les médecines de prévention, notamment la médecine scolaire et la protection maternelle et infantile, doivent être repensées pour faire face aux enjeux actuels, afin « qu'aucun bébé ne naisse prépollué ».

Enfin, certaines mesures pourraient d'ores et déjà, sans attendre les avancées européennes, être mises en place en France pulvériser des produits phytosanitaires, qui sont bien souvent des perturbateurs endocriniens, aux abords des zones d'habitation et des écoles. Les initiatives prises par les professionnels de la petite enfance pour faire des crèches et des lieux de garde des lieux exempts de substances toxiques devraient être encouragées. La formation et la sensibilisation des personnes travaillant au plus près des petits enfants devraient être des priorités. Il ne s'agit pas ici d'hygiénisme ni d'une application exagérée du principe de précaution ; il s'agit plutôt, mes chers collègues, d'encourager l'élaboration d'une véritable politique de santé publique afin d'informer nos concitoyens, de soutenir les initiatives positives en la matière et, surtout, de protéger les générations à venir. La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je remercie le groupe écologiste de nous permettre de débattre aujourd'hui de la lutte contre l'exposition aux perturbateurs endocriniens. d'une question de santé publique essentielle, qui requiert l'action urgente, énergique et concertée des pouvoirs publics nationaux et européens, de la communauté médicale et scientifique, des industriels, des associations et des citoyens. Ces substances omniprésentes dans notre environnement ont fait l'objet d'une définition par l'OMS en 2002 : « Une substance ou un mélange exogène altérant une ou plusieurs fonctions du système endocrinien et provoquant de ce fait des effets néfastes sur la santé de l'organisme intact ou sur celle de sa descendance ». Les perturbateurs endocriniens peuvent agir de différentes façons sur un organisme pour perturber le système hormonal et entraîner des effets néfastes sur la santé imiter une hormone naturelle, bloquer un récepteur hormonal ou modifier les processus de production et de régulation des hormones. Ces modes d'action particuliers permettent de distinguer l'effet endocrinien de l'effet toxique « classique » sur plusieurs points.

plus difficile à détecter. En outre, ce n'est pas la dose qui fait le poison, mais la période d'exposition : le danger est ainsi plus grand pour les femmes enceintes, les enfants de moins de trois ans et les adolescents. Ajoutons que les perturbateurs endocriniens peuvent agir selon une relation dose-réponse non linéaire, ce qui signifie que de faibles doses peuvent avoir des effets plus importants que des doses plus élevées. Enfin, les effets des perturbateurs endocriniens peuvent se transmettre à la descendance. Dans une tribune publiée le 29 novembre dernier, près de cent scientifiques ont alerté l'opinion sur ce danger, dans des termes d'une particulière gravité : « Jamais l'humanité n'a été confrontée à un fardeau aussi important de maladies en lien avec le système hormonal. La très grande majorité des scientifiques activement engagés dans la recherche des causes de ces évolutions préoccupantes s'accordent pour dire que plusieurs facteurs y contribuent, dont les produits chimiques capables d'interférer avec le système hormonal

presque impossible de réduire efficacement l'exposition à ces produits à un niveau individuel. La seule action durablement efficace est donc la réglementation, en amont, de l'utilisation de ces substances, avec pour objectif l'interdiction du recours aux substances identifiées comme perturbateurs endocriniens. Ainsi le bisphénol A, le perturbateur endocrinien le plus connu du grand public, a-t-il été interdit,

élaborée par un groupe de travail réunissant l'ensemble des parties prenantes et adoptée par le Gouvernement en avril 2014. Sa mise en oeuvre constitue l'une des actions phares du troisième plan national santé environnement. Cette stratégie particulièrement ambitieuse et volontariste, qu'il faut saluer, regroupe quatre axes principaux la recherche, la valorisation des travaux et la surveillance des effets des perturbateurs endocriniens ; l'expertise sur les substances ; la formation et l'information des professionnels et du grand public ; l'influence que la France

Ils préconisent également l'interdiction des pulvérisations aux abords des zones d'habitation et des écoles. Il est bon que toutes ces questions soient abordées, même si les solutions simples et radicales sont loin d'être toutes réalisables à court terme- nous y reviendrons. beaucoup question des perturbateurs endocriniens ces dernières semaines, dans le cadre de la campagne électorale, notamment. Je souhaite pour ma part

endocriniens, adopté par la commission des affaires européennes le 12 janvier dernier, ainsi qu'une proposition de résolution européenne adoptée à l'unanimité. Permettez-moi, mes chers collègues, de profiter de ce débat pour pour rappeler les principales conclusions de nos travaux et pour encourager le Gouvernement, déjà expressément engagé en la matière, à déployer tous les moyens mobilisables pour que la réglementation européenne présente et future applique sans attendre le principe de précaution avec la plus grande fermeté. Il n'existe pas de définition européenne des critères permettant de déterminer si une substance est ou non un perturbateur endocrinien. Les règlements européens encadrant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des biocides prévoient une évaluation de toutes les substances entrant dans entrant dans leur composition et organisent le refus d'autorisation pour les substances identifiées comme perturbateurs endocriniens. Néanmoins, ces deux règlements ne donnent pas de critères permettant de définir un perturbateur endocrinien. La Commission européenne devait proposer une définition au plus tard en 2013, ce qu'elle n'a pas fait conduit à la condamnation de la Commission par le tribunal de l'Union européenne le 16 décembre 2015. La Commission a enfin proposé, le 15 juin 2016, deux projets de textes,

à proposer de critères d'identification pour d'autres produits. Nous ne pouvons que déplorer que cette approche morcelée continue de prévaloir, alors qu'une réglementation globale relative aux perturbateurs endocriniens,

avec certitude un lien de causalité entre la perturbation endocrinienne et l'effet néfaste sur la santé. Cela tient à plusieurs facteurs, notamment à la lenteur des procédures de reconnaissance internationale des protocoles de recherche, mais aussi à la latence existant entre l'exposition au perturbateur et la manifestation de l'effet néfaste. La proposition actuelle de la Commission n'est pas satisfaisante ; elle ne permettra pas, en effet, l'application du principe de précaution, lequel consiste à interdire,

et perturbateur. J'insiste sur ces deux adjectifs essentiels : perturbateurs « présumés » et lien de causalité « plausible » entre la perturbation endocrinienne et l'effet néfaste sur la santé. Ces termes sont repris de la proposition de résolution européenne adoptée par la commission des affaires européennes. La prochaine réunion des experts de la Commission est annoncée au 28 février prochain qu'en sera-t-il, madame la secrétaire d'État ? Je rappelle que le Parlement et le Conseil ne pourront pas amender les textes de la Commission, mais seulement les adopter ou y mettre leur veto. Avec notre collègue Alain Vasselle, nous suivons la procédure avec grande attention, en maintenant un échange d'information avec les services de la Commission. Madame la secrétaire d'État, je sais que nous pouvons compter sur la détermination détermination du Gouvernement, en cohérence avec la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, pour promouvoir une définition ambitieuse et réellement protectrice. Quel est votre sentiment sur la suite de la procédure ? Parviendrons-nous à la mise en oeuvre du principe de précaution au niveau européen ? Vendredi dernier, dans le cadre du règlement REACH, le comité a reconnu quatre phtalates comme hautement préoccupants, à cause de leurs propriétés perturbatrices endocriniennes pour l'homme. C'est une première ! C'est encourageant, mais il reste à se défaire du discours selon lequel, en matière de perturbateurs endocriniens, cas pour d'autres produits toxiques, il existerait un dosage ou un niveau d'exposition non dangereux. Si cette occasion était par malheur manquée, il serait particulièrement difficile de poursuivre de poursuivre isolément, au sein du marché unique européen, une stratégie française, pourtant légitime, d'interdiction et de réglementation stricte de l'utilisation des perturbateurs endocriniens. Je pense à l'interdiction des phtalates ou encore à l'engagement d'un candidat à la présidence de la République d'interdire en France l'utilisation de ces substances et l'importation des denrées utilisant ces substances interdites. Nous ne pouvons avancer isolés Certes, l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que les principes de libre circulation des marchandises et de non-restriction des importations « ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de [ ...] protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ». Toutefois, une interdiction globale et permanente de toute importation de biens et de marchandises serait-elle conforme au principe de proportionnalité ? ? La bataille des normes au niveau européen doit être une priorité absolue, d'autant que les intérêts des industries sont organisés et puissants.

La mobilisation nationale, européenne et internationale doit être à la hauteur de l'enjeu vertigineux de santé publique

Les règlements européens prévoient que toute substance identifiée comme perturbateur endocrinien sera interdite dans la composition des produits phytopharmaceutiques et des biocides.

La Commission européenne a proposé différents critères. Ils doivent permettre l'identification des perturbateurs endocriniens dans les produits phytopharmaceutiques et les biocides. Ces critères ont été proposés dans le cadre d'un acte d'exécution et d'un acte délégué. Ces procédures limitent la compétence de la Commission à la seule proposition des critères. Or ces critères sont, à nos yeux, bien trop restrictifs. Notre collègue Patricia Schillinger et moi-même avons donc déposé une proposition de résolution européenne pour élargir le champ des substances devant être considérées comme des perturbateurs endocriniens. L'ANSES,

Nous n'avons pas souhaité, quant à nous, que les substances suspectées d'être des perturbateurs endocriniens soient considérées comme telles par la Commission européenne. En effet, cela aurait entraîné leur interdiction, et tel n'est pas ce que préconise l'ANSES

En effet, l'alinéa 14 préconise une interdiction globale des pulvérisations aux abords des crèches et des écoles, sans qu'il soit tenu compte de la nature des produits pulvérisés. Cela me semble excessif et ne correspond pas à une application proportionnée du principe de précaution. En outre, à l'alinéa 15, vous demandez au Gouvernement de lutter contre l'utilisation des substances « suspectées » d'avoir un effet perturbateur endocrinien. Or il faut distinguer, parmi les substances qui perturbent le système endocrinien, celles qui n'ont pas d'effet néfaste sur la santé et celles qui ont un effet néfaste sur la santé.

toutes les substances utilisées dans les produits phytopharmaceutiques et suspectées d'être des perturbateurs endocriniens, la rentabilité globale des exploitations chuterait de 40 %.

même à très faible dose, comme l'a rappelé Patricia Schillinger. Ces perturbateurs ne sont donc pas des substances toxiques, mais des substances à action endocrine. L'utilisation du mot « toxicité » pour les perturbateurs endocriniens me gêne donc ; elle est inappropriée, et je préfère parler de « dangerosité ». Mes chers collègues, nous devons oeuvrer auprès de nos partenaires européens pour aboutir au plus vite à une définition des perturbateurs endocriniens permettant de protéger au mieux la santé de nos concitoyens.

elle est connue ou présumée pour ses effets néfastes sur un organisme sain ou sa progéniture ; elle altère le fonctionnement du système endocrinien ; il

Cette définition devrait s'appliquer à tous les secteurs d'activité, facilitant ainsi l'encadrement de l'utilisation des substances identifiées comme perturbateurs endocriniens. C'est l'objectif vers lequel nous devons tendre pour une application raisonnée du principe de précaution.

à l'inquiétude légitime et croissante d'une majorité de citoyennes et de citoyens, qui se sont d'ailleurs exprimés dans le cadre d'une pétition européenne, constatant que l'influence persistante des lobbies industriels, notamment de l'agroalimentaire, s'exerce au détriment de la santé publique.

les produits pharmaceutiques ou cosmétiques, dans les produits d'entretien, bref, dans tous les produits du quotidien ! S'ils ne sont pas tous des cancérogènes certains ou avérés et s'ils ne forment pas un ensemble uniforme, il n'en demeure pas moins que le principe de précaution doit pouvoir s'appliquer.

finalement proposé aux États membres, le 21 décembre dernier, quelques jours seulement après sa condamnation, une définition comprenant trois critères cumulatifs. de la Commission européenne, les perturbateurs endocriniens doivent donc montrer des effets indésirables sur un organisme sain ou sa progéniture ; ils doivent altérer le fonctionnement du système endocrinien ; enfin, ses effets indésirables doivent être une conséquence du mode d'action endocrinien. L'obligation de satisfaire ces trois critères a été jugée trop restrictive, car le fort niveau de preuve attendu ne sera probablement jamais atteint. Par ailleurs, ces nouveaux critères étaient censés s'appliquer seulement aux pesticides et non aux autres secteurs de l'industrie chimique, comme ceux des emballages plastiques ou des produits cosmétiques et d'hygiène, la Commission se permettant d'introduire à cet effet une dérogation. Constatant qu'elle ne parviendrait pas à faire adopter cette définition par les gouvernements nationaux, la Commission européenne a été contrainte de reporter le vote.

hausse des cas de diabète de type 2, de l'obésité et de l'autisme » ? Les effets d'une exposition constante à de nombreux et différents perturbateurs endocriniens sont en outre démultipliés par cet effet « cocktail ». De surcroît, ces substances agissent par fenêtres d'exposition, périodes pendant lesquelles les personnes y sont plus vulnérables, comme l'enfance ou la grossesse. Enfin, l'effet néfaste peut y compris se manifester sur la descendance de la personne dont l'organisme a subi la perturbation. Face à ces conséquences particulièrement graves pour la santé, mon groupe s'est positionné depuis plusieurs années en faveur d'une priorité des impératifs sanitaires de protection de la santé publique sur les intérêts économiques et d'emploi. d'emploi. En France, depuis l'interdiction du bisphénol A dans les biberons en 2009- Marie-Christine Blandin en a parlé -, la lutte contre les perturbateurs endocriniens fait l'objet d'un relatif politique.

orchestrée par les industriels pour retarder l'adoption par la Commission européenne d'une réglementation plus stricte en la matière. En effet, cette résolution appelle l'Europe à mettre en place un groupe international de scientifiques indépendants et les gouvernements à appliquer le principe de précaution aux perturbateurs endocriniens avérés et aux substances présumées. Quant à la proposition de résolution du groupe écologiste, dont nous débattons aujourd'hui, visant à renforcer la lutte contre l'exposition aux perturbateurs endocriniens,

contre l'exposition massive de la population aux perturbateurs endocriniens, notamment en développant la recherche universitaire et la recherche publique, et en intervenant au niveau européen pour que la définition des perturbateurs endocriniens protège la santé publique et l'environnement. J'y vois là les conditions d'une meilleure protection de la santé publique et j'avais espéré que le Sénat, dans sa grande sagesse, voterait cette résolution, comme va le faire mon groupe, à l'unanimité, dans la continuité de notre engagement contre le bisphénol A depuis 2009. Malheureusement,

Elle suscite, à l'instar des biotechnologies il y a quelques années, des débats passionnés dans la communauté scientifique, environnementaliste et politique. Si l'existence des perturbateurs endocriniens ne fait aucun doute,

du quotidien de l'homme du XXI siècle. Pourtant jamais l'espérance de vie n'a été aussi élevée ; jamais la qualité de vie n'a été aussi bonne.

Les produits phytosanitaires sont eux aussi largement controversés. Là encore, il faut savoir raison garder. Ces substances n'ont pas été inventées

Les méthodes naturelles sont certes séduisantes, mais elles ne sont pas toujours possibles. Des concentrations importantes en métaux lourds sont retrouvées dans des argiles. C'est la preuve que la nature n'est pas toujours aussi douce l'on veut bien nous le faire croire. Quant aux mycotoxines existant naturellement dans certains végétaux en fonction des variations climatiques, sont-elles réellement préférables aux perturbateurs endocriniens ? L'interdiction récente du bisphénol A dans les biberons, les boîtes de conserve et les tickets de caisse a montré que les solutions alternatives ne permettaient pas de faire de miracle : pis, dans cet exemple précis, les produits de substitution candidats disponibles- bisphénol S ou F -se sont révélés au moins aussi toxiques que le bisphénol A et même bien plus persistants que lui dans l'environnement. Le bisphénol F F contient en effet du fluor, le plus puissant des halogènes ! Ainsi, la mention se voulant rassurante pour le consommateur « Ne contient pas de BPA », est désormais devenue un élément d'angoisse lié à la question : « Par quoi le BPA a-t-il été remplacé ? » Cette expérience malheureuse nous montre qu'une interdiction immédiate et globale de ces substances est irréaliste en l'absence de produits de remplacement ayant fait la preuve de leur efficacité et de leur innocuité. Cette collusion entre lanceurs d'alerte médiatisés et une certaine frange du personnel politique à la recherche d'une image de marque positive est une situation bien française, qui ne manque pas de surprendre beaucoup de nos partenaires européens. Pourquoi vouloir à tout prix tracer une frontière entre le monde scientifique et le monde de l'industrie ? Les deux doivent, au contraire, travailler ensemble pour parfaire leurs connaissances respectives et développer une approche pluridisciplinaire, inhérente à ce type de problématique. Notre pays doit apprendre à faire confiance à la science. Il doit aussi apprendre à se méfier des approximations et de la rhétorique « complotiste » des ONG environnementalistes, qui s'en prennent toujours aux intérêts économiques, mais jamais aux intérêts idéologiques. S'il est impératif de dénoncer les « marchands de doute », qui cherchent à nier des risques clairement établis, il faut aussi traquer avec la même rigueur les « marchands de soupçons », qui laissent subsister des inquiétudes contraires aux connaissances scientifiques. Il importe aussi d'établir de meilleures relations entre les différentes agences des États membres. On pourrait imaginer une seule agence européenne dans le domaine environnemental et sanitaire, qui s'appuierait sur une sélection d'experts dans

Quoique ... Il me paraît donc nécessaire de s'appuyer sur une vision européenne et une expertise communautaire, afin d'harmoniser les expertises et d'éviter les distorsions. Il pourrait aussi être intéressant de créer un groupe de travail de type du groupe

Je félicite également nos collègues Patricia Schillinger et Alain Vasselle pour leur excellent rapport d'information fait au nom de la commission des affaires européennes sur la lutte contre l'exposition aux perturbateurs endocriniens. La proposition de résolution européenne a d'ailleurs été adoptée à l'unanimité en janvier dernier. Je les félicite d'autant plus qu'il s'agit ici d'un enjeu de santé publique devant dépasser tout clivage politique. Le sujet est complexe, il nous concerne tous et représente une menace pour la santé. Bien des choses ont déjà été dites. la santé. Bien des choses ont déjà été dites. Les perturbateurs endocriniens sont en effet des substances chimiques, naturelles ou artificielles, qui affectent le fonctionnement du système hormonal et sont responsables du développement de nombreuses maladies, comme certains cancers, l'infertilité ou encore le diabète et l'obésité. Ces substances sont d'autant plus dangereuses qu'il est difficile de s'en prémunir. Ces substances chimiques sont utilisées dans de nombreux produits comme les phytopharmaceutiques ou les cosmétiques. Elles sont également présentes inévitablement dans l'alimentation, dans l'eau potable ou dans l'air. L'utilisation des perturbateurs endocriniens est massive dans tous les secteurs d'activité et elle ne diminue pas malgré les alertes scientifiques très nombreuses insistant depuis des années sur leurs dangers pour la santé humaine. Les scientifiques admettent désormais que, dans certains cas, les substances perturbant le système endocrinien n'agissent pas comme des substances toxiques classiques. La réglementation européenne ne précise pas les critères scientifiques permettant d'identifier ce qu'est un perturbateur endocrinien. Elle prévoyait que la Commission européenne les détermine avant le 14 décembre 2013, ce qui n'a pas été Le tribunal de l'Union européenne a donc condamné la Commission, qui a finalement présenté ses critères d'identification le 15 juin 2016. Pour être identifiée comme perturbateur endocrinien selon la Commission européenne, une substance doit remplir les trois conditions suivantes elle montre des effets indésirables sur un organisme sain ou sa progéniture ; elle altère le fonctionnement du système endocrinien ; enfin, ses effets indésirables sont une conséquence du mode d'action endocrinien. le rapport d'information de mes collègues de la commission des affaires européennes et cette proposition de résolution, le Sénat fait irruption dans le débat sur les perturbateurs endocriniens et vient l'enrichir, comme à son habitude. Mme Archimbaud propose une définition des perturbateurs endocriniens dans les produits phytopharmaceutiques et biocides plus large que celle soumise par la Commission européenne en interdisant non seulement les perturbateurs endocriniens « avérés », mais aussi ceux qui sont « présumés », au nom de l'application du principe de précaution.

En France, le débat autour des perturbateurs endocriniens n'est pas fréquent, mais il reste régulier. En 2015, notre pays avait déjà pris des mesures contre ces perturbateurs, notamment en ajoutant le bisphénol A, présent dans certains emballages, à la liste des perturbateurs endocriniens interdits. Il est plus que nécessaire d'investir davantage dans la recherche pour permettre d'identifier les substances présentant un danger. Ce doit être un thème prioritaire dans le cadre des programmes de recherche européens. Je salue, par ailleurs, la proposition de la commission des affaires européennes de créer un groupe international de scientifiques indépendants et de haut niveau, qui sera capable de fournir une information objective sur ce sujet. Enfin, il me paraît essentiel de bien réfléchir à la notion de perturbateurs endocriniens « suspectés » de faire peser un risque sur la santé. Cette catégorie aurait un impact extrêmement néfaste

Les conséquences concrètes seraient une baisse de 30 % à 40 % du rendement en pommes de terre et en betteraves, par exemple, due au retrait de certaines molécules. En contrepartie, il serait obligatoire de développer des molécules de substitution qui, selon les industriels, sont estimées à 250 millions d'euros l'unité. Cette proposition de résolution de notre collège Aline Archimbaud vise à prévoir que le Gouvernement renforce son action contre les perturbateurs endocriniens et à faire de la lutte contre l'exposition des enfants aux perturbateurs endocriniens, notamment dans les crèches et les écoles, une priorité de l'action publique. tend à interdire la pulvérisation de produits chimiques, notamment les produits phytosanitaires, aux abords des zones d'habitation et des écoles. Si elle prévoit que la France poursuive son action sur le plan européen ou sur le plan national, en revanche, elle va beaucoup plus loin que des positions de principes.

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je remercie Aline Archimbaud d'avoir déposé cette proposition de résolution visant à lutter contre l'exposition aux perturbateurs endocriniens, qui constituent un enjeu majeur de santé publique, comme vous l'avez tous rappelé avant moi. Je connais l'engagement d'Aline Archimbaud sur ce sujet, comme sur l'ensemble des questions relatives à la santé environnementale. Il s'agit d'un engagement ancien, constant et toujours constructif. Malgré son absence aujourd'hui, je tenais à saluer son travail. Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques dangereuses, très présentes dans notre environnement quotidien. On peut les retrouver dans les produits ménagers, les matières plastiques, les cosmétiques, les textiles, les produits alimentaires ou les jouets.

Les perturbateurs endocriniens sont liés à l'apparition de certains cancers, de l'infertilité, du diabète, de l'obésité ou encore de troubles de développement du cerveau. Ils agissent différemment des autres produits chimiques dangereux, en venant perturber le système hormonal. Ils peuvent interférer avec le système hormonal des êtres vivants à des doses infimes, contrairement aux contaminants plus classiques. Le moment de l'exposition est important, les femmes enceintes et les enfants sont particulièrement sensibles. Les effets peuvent apparaître de façon différée par rapport à l'exposition. Ainsi, les maladies de l'adulte trouvent leur origine dans la période foetale. Les effets sanitaires des perturbateurs endocriniens peuvent être transgénérationnels. la toxicité des perturbateurs endocriniens s'exerce aussi sur la faune sauvage, en particulier aquatique, avec des effets graves sur la capacité de reproduction de nombreuses espèces. Les perturbateurs endocriniens menacent donc la préservation de la biodiversité et la santé des écosystèmes. C'est un sujet C'est un sujet sur lequel je suis particulièrement vigilante, compte tenu de mes responsabilités gouvernementales. Les coûts estimés des perturbateurs endocriniens sur le système de santé européen sont considérables, chiffrés à plus de 150 milliards d'euros par an, représentant plus de 1 % du PIB de l'Union européenne. Il s'agit donc d'un enjeu de santé publique et environnementale majeur, pour lequel le Gouvernement s'est fortement mobilisé. Je salue à ce titre les récentes initiatives sénatoriales, comme la proposition de résolution soutenue par Patricia Schillinger et Alain Vasselle, qui viennent confirmer cette action. La stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens a été mise en place dès avril 2014 par la ministre de l'environnement. Cette stratégie française est une première mondiale et mobilise tous les leviers d'action le levier de la recherche, avec des financements dédiés, et la mise en place d'un programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens ; le levier de l'expertise, avec la mobilisation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement, et du travail, l'ANSES, et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM. Leur travail porte, notamment, sur les substances suspectées d'être des perturbateurs endocriniens et doit permettre de mettre en oeuvre des actions adaptées. Les ministres de l'environnement et de la santé viennent d'ailleurs de saisir l'ANSES sur les substances à expertiser en 2017. Nous souhaitons que l'ANSM poursuive son travail en ce qui concerne les médicaments. le levier de la demande systématique auprès des autorités européennes de mettre fin à la mise sur le marché des substances dès lors que le caractère perturbateur endocrinien est présumé ou avéré ; l'enjeu actuel est d'obtenir une définition satisfaisante et conforme aux avis des experts de la part de la Commission européenne.

Le Gouvernement a également entrepris des actions fortes sur le bisphénol A. Cette substance est utilisée depuis des dizaines d'années pour la fabrication de plastiques, de boîtes de conserve, la vaisselle, les tickets de caisse ou les facturettes de carte bancaire.

L'exposition des femmes enceintes et des jeunes enfants est particulièrement critique, avec des effets différés après l'exposition. À la demande de Ségolène Royal, et grâce à l'expertise de l'ANSES, la Commission européenne a interdit en décembre 2016 l'usage du bisphénol A dans les papiers thermiques, c'est-à-dire les tickets de caisse et facturettes de carte bancaire, car le contact régulier avec les mains des salariées enceintes générait une exposition suffisante pour créer des effets sanitaires sur les foetus. Nous restons néanmoins vigilants quant à l'innocuité des substituts. Le bisphénol S, notamment, fait l'objet de beaucoup d'inquiétudes. À la demande du Gouvernement, la Commission européenne a ainsi chargé l'Agence européenne des produits chimiques de préparer un dossier pour une interdiction, à l'instar du bisphénol A. C'est déjà la France qui avait eu l'initiative d'interdire l'utilisation du bisphénol A dans les biberons il y a quelques années, interdiction reprise au niveau européen. Enfin, depuis le vote de la proposition de loi du député Gérard Bapt, l'utilisation du bisphénol A est interdite dans tous les emballages alimentaires- boîtes de conserve, barquettes plastiques, canettes, etc. -depuis le 1 janvier 2015. La Commission européenne réfléchit à une mesure similaire, mais préfère à ce stade réduire la quantité autorisée dans chaque emballage. Le Parlement européen a voté le 6 octobre dernier, à une très forte majorité, une résolution demandant à la Commission européenne d'aller plus loin, jusqu'à l'interdiction complète comme en France. système de santé a également prévu une réduction drastique de la quantité de bisphénol A autorisée dans les jouets avec pour objectif sa disparition complète. Les ministres Ségolène Royal et Marisol Touraine ont d'ailleurs signé la semaine dernière un projet d'arrêté en ce sens. Dès que Michel Sapin l'aura signé, il sera applicable et le bisphénol A sera enfin interdit dans les jouets en France. Par ailleurs, il est très important de soutenir il est très important de soutenir la recherche sur les perturbateurs endocriniens, afin de pouvoir les identifier précisément. Très bien ! Un appel à projets a été lancé en 2013, le programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens, de même qu'un colloque international a été organisé en 2015. La ministre de l'environnement a mobilisé des fonds du plan Écophyto destiné à réduire l'usage des pesticides. La résolution sénatoriale qui a été votée vendredi dernier, comme la résolution qui est proposée aujourd'hui, vise à demander au Gouvernement de continuer à financer la recherche sur ce sujet. Il est en effet fondamental de soutenir la recherche sur les perturbateurs endocriniens, afin de pouvoir les identifier précisément et de disposer des connaissances scientifiques permettant aux décideurs politiques d'agir et à la population d'être sensibilisée. La stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, la SNPE, a ainsi soutenu le programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens, avec un appel à projets de 750 000 euros en 2013, avec l'organisation de colloques internationaux en France, avec l'expertise importante de l'ANSES portant sur cinq substances par an, dont le BHA et BHT, qui sont cités dans un article du dernier numéro du magazine, et avec la et avec la mobilisation d'un million d'euros le plan Écophyto en 2016. Ces financements ont permis de structurer des équipes de recherche dédiées à ce sujet En ce qui concerne le niveau européen, grâce à notre action et à nos contacts réguliers avec le président de la Commission européenne et des ministres de l'environnement européens, quatre phtalates ont été identifiés le 16 février dernier comme substances chimiques extrêmement extrêmement préoccupantes en raison de leurs propriétés de perturbateurs endocriniens pour l'homme selon le règlement européen REACH. C'est une première, et cette reconnaissance réglementaire permet enfin de mettre en oeuvre les interdictions qui s'imposent. La France vient de déposer un dossier pour que le bisphénol A soit également reconnu au titre du règlement REACH comme perturbateur endocrinien pour la santé humaine. Je sais qu'il y aura des oppositions de la part des industriels, mais cette reconnaissance réglementaire est indispensable pour éliminer cette substance dangereuse. De manière générale, les intérêts particuliers doivent être dépassés pour ériger la santé environnementale au rang de priorité absolue, comme cela aurait toujours dû être le cas. L'outil réglementaire est un volet prioritaire de la stratégie nationale. Vous connaissez l'engagement du Gouvernement au niveau européen pour que les pesticides perturbateurs endocriniens puissent réellement être exclus du marché, ainsi que le prévoit la réglementation communautaire.

Or, il faut le dire, l'attitude de la Commission européenne sur les perturbateurs endocriniens a été décevante. Elle a beaucoup retardé son action, car elle devait modifier la législation sur les pesticides pour le mois de décembre 2013 au plus tard elle n'a présenté un projet qu'au début de 2016, après une condamnation par la Cour de justice de l'Union européenne, à laquelle la France s'était associée. En outre, les règles proposées pour qualifier une substance de perturbateur endocrinien et l'interdire sont très limitatives. Il sera très difficile de proscrire des substances, sauf à attendre que celles-ci aient causé des ravages importants au sein des populations. Le projet de la Commission ne permet pas de prendre en compte les indices et signaux d'alarme précoces. La France s'est beaucoup mobilisée pour faire évoluer la proposition de la Commission européenne, qui, sur ce sujet, doit être plus allante. En effet, notre pays défend une position ambitieuse sur la définition des perturbateurs endocriniens, afin de pouvoir obtenir l'exclusion des substances perturbatrices endocriniennes dans les pesticides et les produits biocides. La France demande ainsi de prendre en compte non seulement les substances perturbatrices endocriniennes avérées, mais aussi présumées, comme c'est le cas pour les substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Par ailleurs, la Commission européenne demande à maintenir sur le marché certaines substances. La France considère que cette dérogation ne peut s'appliquer qu'à des substances pour lesquelles les effets sur les espèces non-cibles sont suffisamment faibles pour ne pas avoir d'impact sur la biodiversité en général, comme les phéromones, qui sont des produits de biocontrôle. Je salue une fois encore la résolution sénatoriale votée vendredi dernier, portée par des sénateurs de sensibilités différentes, ce qui montre que l'intérêt général prime lorsqu'il s'agit de santé et d'environnement. Pas seulement ! La résolution conforte la position française décidée lors de la stratégie nationale, qui est également celle des scientifiques, des experts, ou encore du Parlement européen. Désormais, il est temps que l'Europe se dote d'une réglementation transverse pour réglementer les perturbateurs endocriniens dans les jouets, les cosmétiques, etc. messieurs les sénateurs, des discussions sont en cours entre les ministères et les parties prenantes concernant les épandages de pesticides à proximité des habitations. La ministre de l'environnement a transmis des instructions en 2016 aux préfets pour les arrêtés préfectoraux concernant la nécessité de protéger la population des zones d'épandage à proximité des écoles et des hôpitaux. Soixante-dix arrêtés ont déjà été pris par les préfets. Je partage l'idée, développée dans votre proposition de résolution, qu'il puisse y avoir également des règles claires concernant les zones de non-traitement à proximité des habitations. Je rappelle d'ailleurs que, depuis 1 janvier 2016, les autorisations de mise sur le marché des pesticides peuvent comprendre de telles distances lorsque l'ANSES atteste de leur dangerosité. La mise en place de ces zones de non-traitement est cohérente avec les actions que le Gouvernement a menées, qui s'appuient notamment sur les connaissances scientifiques montrant les effets néfastes des pesticides pour la population et l'environnement interdiction des pesticides pour les jardiniers amateurs en 2019 ; interdiction de la vente en libre-service des pesticides pour le grand public dès cette année ; interdiction des pesticides pour les collectivités dès cette année. Depuis cette semaine, un guide de solutions pour les collectivités qui renoncent à l'utilisation des pesticides fait l'objet d'une large campagne de communication relayée par la presse régionale et nationale.

Le scrutin est ouvert.

La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement. En conséquence, ces candidatures sont ratifiées, et je proclame M. Jérôme Bignon membre du conseil de surveillance, et M. Jacques

Monsieur le président, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, l'eau comme source de vie, l'eau comme bien collectif, l'eau comme droit individuel, l'eau comme objet économique, nécessitant des dispositions singulières : telles sont les bases de la proposition de loi que vous examinez aujourd'hui. Je tiens tout d'abord, au nom du Gouvernement, à saluer la démarche de coconstruction de la proposition de loi La coconstruction s'est d'abord faite avec de nombreuses associations et organisations non gouvernementales humanitaires, caritatives et environnementales regroupées autour d'une plateforme coordonnée coordonnée par la fondation France Libertés et la Coalition Eau. C'est la preuve que nos institutions peuvent pleinement fonctionner en lien avec la société et ses forces vives, et c'est la richesse de notre procédure parlementaire que de permettre à des démarches citoyennes de cette nature de nourrir la discussion dans les hémicycles et d'être examinées par la représentation nationale. Cette coconstruction a également été transpartisane, ce qui n'a rien d'un hasard, car ce texte satisfait un besoin réel de la société française et répond aux difficultés concrètes que connaissent nos concitoyens les plus fragiles et les plus modestes en matière d'accès à l'eau. Introduire dans la loi un droit d'accès à l'eau potable et à l'assainissement peut sembler superfétatoire, tant celui-ci relève de l'évidence pour l'immense majorité de nos concitoyens. Toutefois, c'est oublier la réalité que vivent des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants qui, aujourd'hui encore, sont privés de ces droits qui semblent acquis au plus grand nombre, parce que leur mode de vie n'est pas sédentaire, parce qu'ils vivent éloignés des réseaux, disposent de ressources trop contraintes ou ont perdu leur toit. Ce droit garanti, les conditions de sa mise en oeuvre et de son financement seront au coeur de la discussion parlementaire. Le Gouvernement sera présent pour accompagner vos réflexions et vos orientations, dans le respect de l'initiative parlementaire qui caractérise le texte. Celui-ci prévoit la mise à disposition par les collectivités locales d'équipements sanitaires et d'accès à l'eau potable pour les personnes non raccordées. La décentralisation, c'est la liberté des territoires de déterminer les conditions les plus adaptées à la réalité de chacun d'entre eux pour garantir l'égal exercice des droits. Cette proposition de loi s'inscrit dans cette exigence. Bains douches municipaux, équipements spécifiques dans les centres sociaux chaque collectivité doit avoir le choix des solutions, pourvu que le droit des plus démunis à accéder facilement et sans excès de démarches à l'eau potable et à des équipements sanitaires indispensables à leur dignité leur soit garanti. Inscrire cette exigence dans la loi permet également d'aider les élus locaux qui se heurteraient à des oppositions à la réalisation de tels équipements. Nous savons tous qu'il est difficile de développer des projets de ce type, car ils suscitent d'abord bien souvent- trop souvent -des réticences de voisinage et alimentent parfois des fantasmes. En faire une disposition législative permet aussi d'aider les maires. Le Gouvernement s'est engagé sur ce point à faire adopter une nouvelle tarification progressive de l'eau, de l'électricité et du gaz, afin de garantir l'accès de tous à ces biens essentiels et d'inciter à une consommation responsable. En matière d'énergie, cet engagement est tenu. Plusieurs dispositions de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ont mis en place la traduction concrète de ces principes, notamment au moyen du chèque énergie. En ce qui concerne l'accès à l'eau et sa tarification sociale, « loi Brottes », que vous avez adoptée en 2013, a ouvert aux collectivités locales la possibilité d'expérimenter pendant cinq ans de nouvelles tarifications de l'eau et/ou de l'assainissement, ainsi que des systèmes d'aides au paiement de la facture d'eau, afin de garantir un meilleur accès de tous à ces services. Les dispositifs d'aide aux ménages ayant des difficultés à payer leurs factures d'eau sont ainsi complétés par un volet préventif, car cette expérimentation prévoyait une tarification sociale progressive prenant en compte la situation concrète des ménages, c'est-à-dire leurs revenus et le nombre de personnes composant le foyer. Je salue ici les cinquante collectivités locales qui se sont engagées dans cette expérimentation, laquelle doit permettre de tirer les enseignements des différents dispositifs d'aide, de leur coût de gestion, de leur appropriation par les personnes auxquelles ils sont destinés. Comme les collectivités expérimentatrices elles-mêmes en ont exprimé le souhait, des amendements visent à faire en sorte que cette expérimentation soit prolongée, afin de tester la robustesse dans le temps des dispositifs d'aide, notamment au regard des mises à jour de fichiers. Le Gouvernement aura, sur ces questions, une approche pragmatique. Cette proposition de loi tend à définir non seulement un cadre universel ne reposant pas sur la seule volonté des collectivités, mais aussi une démarche répondant plus vite et de façon générale à la question. Cela suppose de préciser les conditions de la création de l'aide forfaitaire préventive pour l'eau prévue dans la présente proposition de loi. de cette allocation forfaitaire nécessite de définir avec les acteurs concernés des modalités de mise en oeuvre pour s'assurer de son caractère opérationnel et juste, ainsi que pour préciser son financement.

Le Gouvernement souhaite que les débats se poursuivent. Vous le trouverez, au cours de ce débat, attentif, partenaire de cette démarche et disposé à trouver avec vous les meilleures solutions pour garantir la solidarité avec les ménages les plus modestes en matière d'accès à l'eau. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un élément vital, indissociable de la dignité humaine. Je voudrais tout d'abord rappeler que vivre dans une société où l'accès à l'eau n'est pas permis au plus grand nombre est très difficile, et qu'il s'agit toujours d'un enjeu majeur de développement pour les pays dont une partie de la population est privée d'un accès à une eau salubre et à des installations sanitaires. Il suffit de rappeler ce chiffre alarmant : près de 700 000 enfants de moins de cinq ans meurent chaque année du fait de maladies liées à la consommation d'une eau contaminée. En France, le droit à l'eau potable et à l'assainissement est une réalité pour la grande majorité de la population. C'est une chance. 99 % des personnes sont aujourd'hui raccordées à un réseau de distribution d'eau. Pourtant, certaines catégories de population n'ont toujours pas, dans notre pays, au XXI siècle, d'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans des conditions satisfaisantes. Il s'agit, d'une part, des personnes qui n'ont pas d'accès physique à l'eau, notamment les sans-abri, et, d'autre part, de personnes en difficulté qui ont du mal à régler leurs factures d'eau et font face à des impayés, voire à des coupures d'eau.

Ces craintes, je le dis avec force, sont totalement infondées si l'on regarde en détail les mesures que ce texte contient, au-delà de tout fantasme et de toute posture. Exact ! Que prévoit-il ? Premièrement, il inscrit dans la loi la reconnaissance d'un droit à l'eau potable et à l'assainissement. J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de créer un droit opposable, puisque la proposition de loi ne définit pas de voies de recours juridictionnelles pour contraindre la puissance publique à agir. Il s'agit simplement d'inscrire dans Il s'agit simplement d'inscrire dans l'ordre juridique interne un droit qui a été reconnu au niveau international, notamment par la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 28 juillet 2010, dont l'adoption a été soutenue par la France.

Deuxièmement, ce texte prévoit que les collectivités compétentes en matière d'eau et d'assainissement installent et entretiennent des équipements de distribution gratuite d'eau potable. Il prévoit également la mise à disposition gratuite de toilettes publiques dans les collectivités de plus de 3 500 habitants et de douches publiques dans les collectivités de plus de 15 000 habitants, afin, notamment, que les personnes sans-abri puissent satisfaire leurs besoins élémentaires d'alimentation et d'hygiène. Cette mesure est bien loin d'être aussi contraignante qu'il y paraît ou qu'on le dit. Le texte indique clairement que, pour se conformer à ces obligations, les collectivités pourront utiliser des équipements sanitaires existants dans des bâtiments publics, par exemple les vestiaires des centres sportifs, ou dans des bâtiments appartenant à des associations qu'elles subventionnent. Pouvez-vous me citer une commune en France qui ne dispose pas aujourd'hui d'un point d'eau pouvant être mis à disposition des personnes démunies ? Cela n'existe pas

à l'eau, versée sous condition de ressources aux personnes qui ont des difficultés à régler leurs factures d'eau. Cette aide serait attribuée aux personnes dont les revenus sont compris entre le montant du RSA socle et le plafond de ressources de la CMU-C, en intégrant les écarts de prix de l'eau suivant les territoires- c'est une donnée importante.

Une autre objection m'a été faite : pourquoi créer une telle aide alors que les centres communaux d'action sociale, les CCAS, et les fonds de solidarité pour le logement, les FSL, gérés par les départements, accordent déjà des aides aux ménages en difficulté pour régler leurs factures d'eau.

Nous sommes très nombreux ici à nous alarmer de l'incapacité des départements à assumer la totalité de leurs compétences d'action sociale.

J'en viens maintenant à la question du financement de cette aide. Le Conseil général de l'environnement et du développement durable, le CGEDD, a estimé le coût d'une telle aide entre 50 et 60 millions d'euros, à comparer avec le chèque énergie, dont le coût est de l'ordre de 600 millions d'euros. Dans sa version initiale, la proposition de loi prévoyait la création d'une taxe additionnelle à la taxe existante sur l'eau en bouteille de 0,5 centime d'euro par litre. Cela représentait globalement 1 euro par an et par consommateur d'eau en bouteille, ce qui n'était pas une somme considérable Cette surtaxe a été supprimée par l'Assemblée nationale, sur l'initiative du Gouvernement et de plusieurs députés. Désormais, il est prévu que cette aide soit financée par la taxe existante sur l'eau embouteillée, qui est affectée

nationale. Enfin, la proposition de loi prévoit de mobiliser les collectivités sur le suivi de la mise en oeuvre du droit à l'eau potable et à l'assainissement par l'organisation d'un débat sur les actions prévues ou menées en la matière dans les trois ans suivant les élections municipales. Vous le voyez, mes chers collègues, cette proposition de loi répond à l'enjeu majeur de l'accès à l'eau en mettant en place un dispositif simple et peu coûteux d'aide sociale. Voilà des années que la question du droit à l'eau et de la création d'une aide préventive est débattue. Ce texte s'inscrit dans le cadre des nombreux travaux qui ont été conduits sur cette question par des juristes, des associations, ou encore par le Comité national de l'eau et le Conseil d'État. temps d'aboutir et de faire du droit à l'eau potable et à l'assainissement une réalité partagée par tous. Telle est l'ambition de cette proposition de loi. Elle a été signée et votée par des députés de quatre groupes politiques différents, pas seulement de gauche, à l'Assemblée nationale. J'espère que le Sénat,

le présent texte aborde une question fondamentale, celle du droit à l'eau. Toutefois, comme l'a très bien dit notre rapporteur, Ronan Dantec, dont je salue au passage l'excellence du travail et la force de conviction, il ne fait pas que proclamer ce droit. Il lui donne corps par deux mesures concrètes. La première est l'obligation pour les collectivités locales, singulièrement les communes et les EPCI, de fournir à toute personne qui en serait dépourvue un point d'accès à l'eau pour ses besoins élémentaires. La seconde mesure de concrétisation du droit à l'eau est la création d'une allocation forfaitaire permettant aux ménages les plus nécessiteux de s'acquitter de leur facture d'eau. Néanmoins, sur qui va peser la mise en oeuvre du droit à l'eau ? Sur les collectivités locales ! C'est bien là que le bât blesse. Pas du tout, nous rétorque Ronan Dantec, aucune charge nouvelle ne pèsera sur les collectivités. Au contraire, elles en bénéficieront. Premier argument : ne craignez rien, il ne s'agit pas d'un droit opposable. Deuxième argument : l'obligation de garantir un accès à l'eau potable, à des toilettes, des douches et des laveries ne pèsera pas sur les collectivités parce qu'elle est déjà satisfaite. qu'elle est déjà satisfaite. Toutes les communes visées par le texte disposeraient déjà des infrastructures concernées. Le droit à l'accès à l'eau serait donc effectif. Troisième argument : les collectivités bénéficieraient de l'instauration de l'allocation forfaitaire d'eau.

son fonds de solidarité pour le logement, le FSL, lorsque la consommation d'eau est facturée dans les charges du logement, soit sur la commune, le centre communal d'action sociale, ou CCAS, lorsque la facture d'eau est individualisée. Or, en créant une aide préventive, le présent texte en assure le financement par l'État. L'allocation forfaitaire d'eau sera en effet financée par la taxe sur les eaux en bouteille. Aujourd'hui, cette taxe est intégrée dans le budget général de l'État. Elle serait désormais fléchée vers le Fonds national d'aide au logement, qui la distribuerait aux FSL, lesquels auraient l'obligation de créer un fonds « eau » en leur sein. Le produit de cette taxe est de 50 à 60 millions d'euros. Les besoins estimés de l'allocation forfaitaire d'eau sont du même montant. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes ! L'idée est que l'instauration de l'allocation forfaitaire préventive assèche les besoins d'aides curatives. Par conséquent, le gain pour les collectivités de la création de l'allocation forfaitaire d'eau ne serait pas seulement financier : ce serait aussi un gain de gestion. Malheureusement, ces arguments ne sont pas convaincants. Celui de la non-opposabilité du droit à l'eau est bien curieux pour qui prétend concrétiser un véritable droit. Cela revient à dire que, si le droit à l'eau emporte des obligations de la part de la collectivité, elles ne seront pas sanctionnées. En quoi ce droit n'est-il pas alors simplement déclaratif ? De plus, pourquoi le droit nouveau ne serait-il pas opposable ? À partir du moment où il sera inscrit dans la loi, rien n'interdira d'intenter des recours sur son fondement. L'argument selon lequel ce texte ne modifiera rien pour les collectivités parce qu'elles fournissent déjà un service d'accès à l'eau interroge sur l'utilité du texte. Qu'apporte-t-il s'il ne change rien ?

D'ailleurs, aucun élément chiffré n'est produit à l'appui de cette affirmation. Les communes de plus de 3 500 habitants disposent-elles toutes de toilettes publiques et de points d'eau potable accessibles à tous ? Celles de plus de 15 000 habitants proposent-elles toutes des douches et des laveries gratuites Nous n'en savons rien, puisque le présent texte est une proposition de loi et que, par conséquent, il n'est pas accompagné d'une étude d'impact. Si le droit à l'eau est si fondamental, pourquoi ne pas avoir présenté un projet de loi associé à une étude d'impact ? Le texte lui-même contredit l'idée que toutes les installations existeraient déjà, puisque son article 2 prévoit que les collectivités de plus de 15 000 habitants « installent » des douches gratuites, ce qui indique bien qu'elles n'en disposent probablement pas toutes. Surtout, disposer des infrastructures et les mettre à disposition sont deux choses bien différentes ! En effet, même si les infrastructures existent, cela coûte de les rendre accessibles, en termes d'exigences de sécurité et, encore plus sûrement, d'entretien. Les représentants des collectivités que nous sommes ne peuvent qu'être sensibles à ces charges sans cesse accrues et jamais compensées. Il est du devoir de la Haute Assemblée de dire : « Stop ! ». Quant à l'argument invoqué à l'appui de la création de l'allocation forfaitaire d'eau, il n'est pas non plus totalement convaincant, pour au moins deux raisons. La première, c'est que rien ne garantit qu'elle « siphonne » effectivement les besoins actuels en aide curative. La seconde est que la gestion du dispositif continuera d'incomber aux collectivités. Le texte ne prévoit pas autre chose. Il y est même écrit le contraire à l'article 4, qui prévoit un rapport relatif à « l'opportunité de rapprocher le dispositif de l'allocation forfaitaire d'eau du dispositif du chèque énergie En attendant, ce seront bien toujours aux collectivités d'instruire et de gérer les dossiers. Par ailleurs, il y a deux points importants sur lesquels le texte demeure totalement muet. Le premier est celui de son application outre-mer. Aucune modalité d'application différenciée n'est prévue, alors qu'elle s'imposerait à l'évidence. Le second point clef ignoré par la proposition de loi est celui de l'éducation à l'usage de l'eau. La concrétisation du droit à l'eau emporte en effet le risque de faire passer l'eau pour quelque chose de gratuit,

conclure, si le présent texte aborde une question fondamentale et y apporte un début de réponse, il comporte encore de trop importantes zones d'ombre concrètes et techniques. D'un point de vue strictement législatif, dans sa mouture actuelle, il n'est pas abouti, ne serait-ce que parce que les charges qu'il crée pour les collectivités ne sont pas assumées, ni financièrement ni politiquement.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, comme l'a excellemment souligné notre rapporteur Ronan Dantec, que je remercie chaleureusement, la proposition de loi que nous examinons cet après-midi est l'aboutissement d'un long travail de réflexion et de négociation avec de nombreuses ONG, parmi lesquelles la fondation France Libertés a joué un rôle essentiel. Nous sommes fiers que ce texte, de portée universelle et relatif à la défense des droits humains et des biens communs, ait pu enfin être inscrit à l'ordre du jour du Sénat. Je le rappelle, cette proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale par Michel Lesage et six autres députés

Cette proposition de loi a pour objectif d'inscrire ce droit d'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans le droit français, suivant ainsi la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, qui avait affirmé, le 28 juillet 2010, ce droit d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. N'oublions pas que ce combat pour la reconnaissance du droit à l'eau et à l'accès à l'eau potable a été mené inlassablement par celle qui fut la présidente de la fondation France Libertés, Danielle Mitterrand. Elle a toujours été à l'avant-garde pour démontrer la contradiction entre le statut naturel de l'eau et son exploitation économique, en sensibilisant les citoyens aux dangers de la privatisation de ce bien commun. Comme l'air que l'on respire, l'eau est un bien commun qui ne peut être considéré comme une marchandise. Ce principe est inscrit dans le premier article de la charte des porteurs d'eau- un mouvement international -, qui fait de chaque citoyen « porteur d'eau » un militant pour une gouvernance mondiale de l'eau, pour que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement soit un droit inaliénable pour tous. En juin En juin 2010, nous avions d'ailleurs signé officiellement cette charte des porteurs d'eau à Bordeaux avec la présidente de la fondation France Libertés et le conseil départemental que je présidais. Élément indispensable de la dignité humaine, dénominateur commun à toute forme de vie sur terre, l'eau est devenue un enjeu géopolitique, à l'origine de migrations et de guerres au XXI siècle. Enjeu de solidarité territoriale et de coopération internationale, l'eau se trouve au coeur du changement climatique et de la transition écologique. L'eau est une source de vie, mais, lorsqu'elle vient à manquer, par exemple lors des catastrophes naturelles- on l'a vu récemment lors des tragiques séismes en Haïti ou au Népal en 2015, ou encore à Mayotte -, elle devient la cause de terribles épidémies et de mort. Il est important de rappeler des données chiffrées : 34 000 personnes meurent chaque jour dans le monde par manque d'accès à l'eau potable, dont 5 000 enfants 1,5 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et 2,6 milliards à l'assainissement. Ces données relatives à la situation dans le monde ne doivent pas faire oublier qu'en France, la cinquième puissance économique mondiale, des milliers de personnes ne disposent pas de branchement à l'eau potable ou n'ont pas les ressources suffisantes pour payer cet accès à l'eau. C'est ainsi que notre pays est loin de respecter les recommandations des Nations unies, qui prévoient un minimum indispensable de 20 litres d'eau par personne et par jour. L'un des objectifs de cette proposition de loi est de contraindre les collectivités locales à installer et entretenir des équipements de distribution gratuite d'eau potable, ainsi que la mise à disposition de toilettes publiques dans les communes de plus de 3 500 habitants et des douches publiques dans celles de plus de 15 000. Une telle mesure doit permettre aux sans-abri de satisfaire leurs besoins élémentaires d'hygiène et d'alimentation. En outre, de telles installations existent déjà ; l'effort des communes devra porter uniquement sur la visibilité et l'accès à ces équipements. ce propos, vous me permettrez de souligner le travail qui est actuellement réalisé dans la métropole bordelaise pour raccorder à l'eau potable une cinquantaine de squats. Ces actions, qui concernent environ 1 000 personnes, favorisent la scolarisation des plus jeunes, évitent le risque de maladies à potentiel épidémique, ainsi que la dégradation des biens publics et privés. Une autre mesure symbolique contenue dans ce texte est la création d'une allocation forfaitaire d'eau, qui permettrait de venir en aide aux familles ne pouvant pas payer leurs factures. Cette aide s'adresserait aux personnes dont les dépenses d'eau excèdent 3 % de leurs revenus disponibles et concernerait environ 2 millions de personnes en France. Compte tenu des différences du prix de l'eau sur l'ensemble de notre territoire, cette « allocation solidarité eau » ne serait attribuée qu'aux seules personnes payant l'eau à un prix supérieur au prix fixé par décret. Le coût de cette aide est estimé entre 50 et 60 millions d'euros. Ces mesures, qui tendent à rendre leur dignité à toutes ces populations privées d'eau, sont faciles à mettre en oeuvre, et la plupart d'entre elles viennent compléter les dispositifs déjà existants comme la loi Brottes du 15 avril 2013, qui a permis l'interdiction des coupures d'eau ; les nombreuses et récentes décisions de justice condamnant les entreprises industrielles de l'eau vont d'ailleurs faire jurisprudence. L'obligation qui est faite d'organiser des débats autour de l'eau dans les assemblées délibératives des communes montre que le terrain de l'eau ouvre les portes d'une éducation citoyenne responsable des pratiques démocratiques la tenue de tels débats aura l'avantage de rendre les enjeux de l'eau plus lisibles, avec la prise en compte de la dimension du rôle des usagers. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, vous l'avez bien compris, ce combat mené pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est le symbole emblématique de tout un engagement pour un monde plus juste et plus solidaire ! Après la COP21 et le vote de la loi sur la biodiversité, la France doit montrer l'exemple, en s'engageant encore pour un modèle respectueux de l'environnement, de la ressource en eau, de la promotion des droits humains. Au niveau tant local qu'international, l'eau est un enjeu de gouvernance et la gestion de ce bien commun doit plus que jamais être au service au service des communautés et de l'intérêt général. Mes chers collègues, l'adoption de ce texte constituerait une première étape, un fondement dans la reconnaissance de la dignité humaine : le droit à l'eau pour tous. « L'eau, c'est la vie ! », répétait inlassablement Danielle Mitterrand. L'eau, c'est un droit, un droit inaliénable à inscrire dans la Constitution. Avec ce texte, la France serait pionnière, un modèle pour les autres pays, suivant l'exemple de la Slovénie en Europe, et bien après le Burkina Faso, la Tunisie, l'Afrique du Sud, l'Uruguay, le Venezuela

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes invités par nos collègues écologistes à discuter d'une proposition de loi, adoptée à l'Assemblée nationale, qui vise à mettre en oeuvre le droit à l'eau potable et à l'assainissement. Ce texte a un objectif louable. Malheureusement, je regrette qu'il ne soit pas accompagné des outils nécessaires pour l'atteindre. Pis encore, il contient des dispositions aux portées normatives pour le moins discutables, dont il est impossible de chiffrer les coûts en l'absence d'étude d'impact. Cela commence dès le premier article. Celui-ci comprend le droit pour chaque personne physique de disposer d'une quantité suffisante d'eau potable- difficile de s'y opposer, je vous l'accorde ! Malheureusement, cette mesure pourrait bouleverser l'équilibre qui résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales, le CGCT, sur le service public de l'eau et de l'assainissement. En effet, le CGCT précise que les communes arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. si une construction ne figure pas dans une zone desservie par le réseau de distribution, la commune n'a pas d'obligation de raccordement. Par conséquent, le droit à l'eau potable et à l'assainissement, tel qu'il est prévu dans la proposition

l'installation d'équipements de distribution gratuite d'eau potable, l'installation des toilettes publiques gratuites dans les collectivités de plus de 3 500 habitants et des douches publiques gratuites pour les collectivités de plus de 15 000 habitants. Pouvons-nous réellement nous permettre de solliciter de nouvelles dépenses à la charge des collectivités territoriales, déjà étranglées par les récentes décisions financières ?

En somme, vous demandez aux agences de l'eau de faire plus avec moins : cela n'est pas possible ! Quant aux articles 3 et 4, ils visent l'introduction de deux mécanismes d'aide préventive l'aide préventive pour l'eau, à l'article 3, et la création d'une allocation forfaitaire d'eau pour les ménages les plus pauvres, à l'article 4. Ces dispositions vont déresponsabiliser nos concitoyens. d'abord sur le plan économique : il s'agira d'anticiper des situations d'impayés consécutives, soit du fait d'un prix de l'eau trop important, comme le prévoit le mécanisme d'allocation forfaitaire d'eau prévu à l'article 4, soit du fait de dépenses d'eau trop importantes au regard des ressources des ménages, comme le prévoit l'aide préventive pour l'eau à l'article 3. Ensuite, cela va aussi déresponsabiliser nos concitoyens sur le plan écologique, puisque de tels mécanismes ne peuvent que décourager les comportements vertueux en termes de consommation raisonnée d'eau potable. Enfin, l'absence d'étude d'impact concernant les articles 3 et 4 ne nous permet pas, en tant que législateur, d'appréhender les conséquences économiques et sociales. attaché à la simplification des normes, je ne puisse m'associer à des mesures qui pourraient se traduire par la naissance de nouvelles normes. on nous explique que le produit de la contribution sur les eaux et boissons embouteillées, dont les sommes perçues par la douane sont mises à la disposition de chaque commune concernée, sera fléché vers l'allocation de logement social, qui est une composante du Fonds national d'aide au logement, Néanmoins, cette allocation n'a rien à voir avec l'allocation forfaitaire d'eau, puisque celle-ci est une autre composante du FNAL ... Ainsi, l'article 6 ne permet pas d'apporter de nouvelles sources de financement en faveur de l'aide préventive pour l'eau de l'article 3, ni pour l'allocation forfaitaire d'eau prévue à l'article 4. il n'est nullement mentionné que ces fonds accompagneront les collectivités territoriales dans le financement des nouvelles obligations prévues par l'article 2. Enfin, et peut-être ne l'avez-vous pas vu, monsieur le rapporteur, les dispositions de l'article 6 affecteront négativement le régime vieillesse des non-salariés agricoles.

ne votera pas cette proposition de loi, que je considère pour ma part- pardonnez la franchise de mes propos ! -comme un puits sans fond. Très bien ! La parole est à M. Bernard Vera. Monsieur le

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'effectivité du droit à l'eau est un sujet récurrent dans notre hémicycle. En effet, si la loi sur l'eau et les milieux aquatiques a défini un droit à l'eau à son article 1, aujourd'hui encore aucun instrument légal ne permet réellement de le garantir. Cette absence est contradictoire avec les engagements internationaux pris par la France, notamment dans le cadre de l'ONU. Il convient donc que le législateur donne corps à ce droit fondamental par l'adoption de dispositifs efficaces, ce qui est l'objectif de ce texte. Je rappelle que notre groupe avait déposé, dès 2009, une proposition de loi sur ce sujet. Nous avions d'ailleurs tenté d'insérer ces dispositions lors de la discussion sur les aides versées aux ménages pour faire face aux impayés, une proposition de notre collègue Christian Cambon abordant le volet curatif du droit à l'eau. Absolument ! Nous abordons aujourd'hui l'autre versant de ce droit, le volet préventif, afin de consacrer le droit à l'eau et à l'assainissement comme un droit réel et tangible. Ce long travail de conviction a été mené avec des associations, le Comité national de l'eau, la Coordination eau. Il est maintenant assumé par la fondation France Libertés. Le constat est clair et partagé par tous les acteurs : si l'eau est un bien commun, rare et précieux, son accès doit être garanti à tous dans sa dimension eau potable, par une « allocation eau », ainsi que par un accès à l'assainissement. Cela passe d'abord par de nouvelles obligations incombant aux collectivités en matière sanitaire, par des douches, des toilettes et des points d'eau obligatoires. Un tel dispositif, s'il fait peser des obligations sur les collectivités, apparaît comme nécessaire et justifié au regard de l'importance de cet accès pour la dignité de chacun. Nous y sommes favorables. Concernant l'accès à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables, le programme national des Nations unies indique que l'accès à l'eau ne doit pas dépasser 3 % des ressources d'un ménage. Par cette proposition de loi, il s'agit donc d'organiser une véritable garantie légale d'accès à l'eau. C'est la même recherche qui avait guidé le dépôt de la proposition de loi par notre groupe en 2009. Pour autant, il faut souligner que le contenu était légèrement différent. Nous proposions à l'époque la distribution d'une allocation eau, sur le modèle des APL, une allocation dispensée par les CAF et financée par les distributeurs d'eau taxés à hauteur de 1 % de leur chiffre d'affaires. S'il reste dans cette loi le principe d'une allocation eau, les modalités de versement et les seuils sont laissés à l'appréciation du pouvoir réglementaire. Par ailleurs, la proposition de loi déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale a évolué vers un financement de ce dispositif par une taxation additionnelle sur les eaux embouteillées. Depuis des années, ce volet préventif du droit à l'eau achoppe principalement sur la question du financement, et cette nouvelle proposition voulait faire consensus. Pourtant, l'Assemblée nationale, par l'adoption d'un amendement du Gouvernement et du groupe Les Républicains, a supprimé purement et simplement le financement prévu, fléchant simplement l'actuel produit de la taxe sur les eaux embouteillées vers le financement de l'allocation. Pour ce qui nous concerne, nous n'étions pas opposés par principe à ce type de financement par une taxe additionnelle. Pour autant, le discours selon lequel les consommateurs de bouteilles d'eau peuvent financer ce surplus met totalement de côté le fait même qu'en tout point du territoire la qualité de l'eau n'est pas la même et que certains de nos compatriotes n'ont pas le choix. Une récente étude de l'a d'ailleurs souligné ce point. Par ailleurs, cette source de financement met, encore une fois, les seuls consommateurs à contribution, puisque- nous le savons -cette taxe serait directement répercutée sur le prix de l'eau embouteillée. Quand allons-nous enfin faire contribuer les de l'eau, et non les consommateurs ? Sur le fond, il faut être clair. Ce dispositif d'accompagnement social pour l'accès à un droit fondamental n'est pas, dans notre esprit, un aboutissement, mais un premier pas vers un service public de l'eau. En effet, s'il est important de pallier une inégalité manifeste, il reste fondamental de rappeler que l'eau est un bien commun auquel tout le monde a droit, un bien vital qu'il faut sortir des logiques marchandes. D'ailleurs, de nombreuses collectivités, et non des moindres, ont fait le choix d'un retour en régie publique. Nous craignons malheureusement que les réformes territoriales ne menacent directement les régies existantes par la marche forcée vers des intercommunalités géantes qui ne tiennent pas compte de la géographie et des bassins versants. Nous sommes une fois de plus face à une vision gestionnaire qui tient peu compte de la réalité. Au-delà de la création de cette allocation eau, il convient parallèlement d'aider les collectivités à faire baisser la facture pour l'ensemble des usagers, en posant la question du prix de l'eau, donc celle de la rémunération des gestionnaires des délégations de service public. En effet, les profits dans le secteur de l'eau sont très confortables, ce qui n'est plus acceptable, pas plus d'ailleurs que les poursuites engagées par Veolia contre les dirigeants de France Libertés pour diffamation. Un procès se tiendra le 9 mars prochain et nous espérons que la justice protégera ces personnes, dont le seul tort est de dénoncer la poursuite des coupures d'eau et d'appeler à la vigilance sur les méthodes commerciales agressives de cette société en matière d'avenants aux contrats de délégations. Nous soutenons donc fermement le combat de ces associations. Au-delà de ces considérations, il n'en demeure pas moins que, aujourd'hui, nous avons le choix : celui de marquer ou non un pas vers un droit à l'eau dans des conditions juridiquement garanties et économiquement acceptables. Il serait regrettable que le Sénat balaye d'un revers de main un travail aussi long et minutieux que celui qui a été réalisé par les auteurs de la proposition de loi et par les associations. Pour toutes ces raisons, nous soutiendrons évidemment ce texte, sans proposer de modification, afin qu'il soit adopté de manière conforme, donc définitive, par les deux assemblées. Mes chers collègues, cette proposition de loi apporte une aide concrète et juste à nos concitoyens dans l'exercice d'un droit essentiel reconnu par la loi : le droit à l'eau.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, avec 600 millions de personnes privées d'eau salubre et plus de 2,5 milliards d'individus ne disposant pas d'un accès à des installations sanitaires, le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un enjeu majeur de développement. Face à cette situation, comme cela a été rappelé, ce droit a été inscrit dans différents traités internationaux et il a été reconnu comme fondamental par les Nations unies le 28 juillet 2010. Si cette question concerne bien entendu avant tout les pays en développement, il se trouve encore en France des catégories de population qui n'ont pas facilement accès à l'eau et à l'assainissement : les sans-abri et les personnes pour lesquelles cette charge économique est difficilement supportable. En proposant la mise en oeuvre effective du droit à l'eau potable et à l'assainissement, le texte s'adresse à ces catégories. Son objectif est louable. Comment, en effet, ne pas souscrire au principe de la reconnaissance du droit à l'eau potable et à l'assainissement, comme le prévoit l'article 1 ? L'eau est un bien vital, qui doit être garanti pour tous. Bien entendu, nous ne partons pas de rien. S'il faut reconnaître que la disparition des fontaines publiques et des bains-douches complique la vie des sans-abri, les ménages en difficulté peuvent, en revanche, bénéficier d'un certain nombre de mesures leur permettant de faire face aux impayés ou aux coupures d'eau. Ces aides, comme vous le savez, mes chers collègues, sont mises en oeuvre par les centres communaux d'action sociale ou les fonds de solidarité pour le logement. Les FSL distribueraient ainsi un peu plus de 300 millions d'euros par an, au bénéfice d'environ 600 000 ménages. Citons aussi la loi Brottes, qui prévoit l'interdiction des coupures d'eau en cas d'impayé, une interdiction qui s'exerce tout au long de l'année, ainsi que la possibilité d'expérimenter la tarification sociale. Il est certain que ces dispositifs pourraient être améliorés pour mieux identifier et accompagner les particuliers. Je pense notamment aux FSL, dont un quart ne comporterait pas de volet « eau ».

Par ailleurs, sans nier la nécessité de favoriser l'accès à l'eau et à l'assainissement dans l'espace public, doit-on faire encore une fois peser l'essentiel de l'effort sur les collectivités locales, comme si elles n'en faisaient pas déjà

douches publiques gratuites dans les collectivités de plus de 15 000 habitants -, d'autant que les collectivités territoriales doivent se débattre avec des budgets contraints et des baisses constantes de dotation. N'en rajoutons donc pas, cela pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase Les collectivités locales ont la compétence « eau ». Beaucoup d'entre elles assument leurs responsabilités et mettent en oeuvre des actions de solidarité dans le domaine de l'eau, en particulier en milieu rural, où les besoins sont facilement identifiés. Certes, dans certains territoires, on peut mieux faire, en particulier dans les grandes villes, qui sont les plus concernées par la question des sans-abri. Un effort substantiel d'équipement pour atteindre un ratio suffisant de toilettes publiques par

mettent en oeuvre des politiques de proximité pour tenter de garantir les droits les plus fondamentaux de leurs administrés. C'est la raison pour laquelle le groupe du RDSE ne votera pas en faveur de cette proposition de loi trop contraignante pour les collectivités territoriales, en particulier dans le contexte actuel.

pour son dernier espace réservé, le groupe écologiste a pensé utile de reprendre une proposition de loi transpartisane déposée et adoptée à l'Assemblée nationale, défendue par M. le député Michel Lesage et ayant pour thématique l'eau pour tous. Notre débat porte sur la mise en oeuvre du droit humain à l'eau potable et à l'assainissement. L'effectivité de ce droit est nécessaire pour permettre un égal accès à une ressource vitale à la survie de l'espèce humaine, cela a été suffisamment dit. D'un point de vue tant sanitaire que social, il est urgent et de l'intérêt de tous de permettre cette égalité.

! Dans ce texte, il est proposé de reconnaître en droit français le droit à l'eau potable et à l'assainissement, reconnaissance qui existe déjà à l'échelon international puisque deux résolutions de l'ONU, de 2010 et de 2013, qualifient ce droit de « fondamental ». Il s'agit aussi de garantir un accès physique à l'eau potable et à des équipements sanitaires, créer une aide préventive d'accès à l'eau et à l'assainissement pour les bénéficiaires du RSA socle et d'organiser un débat sur la mise en oeuvre de ce droit.

on ne peut pas avoir comme seule réponse « C'est trop cher, attendons demain que nous soyons plus riches » ! Ce n'est pas possible ! Au-delà des enjeux sociaux et de santé publique, la mise en place d'équipements sanitaires ou de distribution d'eau participe également

L'effectivité du droit à l'eau est également mise à mal par les difficultés que rencontrent certains ménages à payer leur eau. Un consensus existe pour considérer que le coût est excessif lorsque la facture dépasse 3 % des revenus. Or le constat est édifiant environ un million de ménages sont confrontés à une facture excessive et ne seraient donc pas en mesure de la payer. Ce phénomène entraîne des impayés, eux-mêmes à l'origine de coupures d'eau, qui privent des familles de l'accès à cette ressource vitale. Cette situation est inacceptable ! Face à cette réalité, l'association France Libertés et d'autres ont proposé au législateur un certain nombre de modifications du droit afin de prévenir ces difficultés. Tel est l'objet du texte discuté aujourd'hui, qui propose de mettre en place une aide préventive d'accès à l'eau et à l'assainissement. Cette nouvelle aide ne pèsera pas sur les collectivités territoriales. En effet, la présente proposition de loi prévoit l'affectation du produit de l'actuelle contribution sur les eaux embouteillées au financement de cette aide, contrairement à ce que vous disiez, monsieur Pointereau. À terme, cette aide permettra même de diminuer le coût des aides curatives. En effet, les fonds de solidarité pour le logement et les centres communaux d'action sociale auront de moins en moins de coûts de gestion liés aux dossiers d'impayés puisque ces derniers diminueront grâce à l'application de cette loi. de cette loi. La proposition de loi examinée aujourd'hui présente un double avantage : elle reconnaît un droit effectif à l'eau potable et à l'assainissement tout en offrant un cadre juridique souple aux collectivités territoriales, ne vous en déplaise, monsieur Pointereau. Oh ! Encore ? Cette position de compromis ne résulte pas du hasard. Ce texte, porté, je le rappelle, par des députés de quatre groupes politiques différents, a été construit en partenariat avec des associations comme France Libertés et certaines institutions. Soutenu par les embouteilleurs et les services de gestion des eaux, il a évolué pour tenir compte de la position du Gouvernement lors de sa lecture à l'Assemblée nationale. Veuillez conclure, monsieur Desessard

Voilà qui résume parfaitement, en quelques mots, mon propos. Comme le disait le député Michel Lesage, cosignataire de cette proposition de loi particulièrement opportune, « l'eau est bien le reflet de nos communautés humaines.

». Selon la résolution de l'ONU, le droit à l'eau potable et à l'assainissement est bien « un droit fondamental, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme Il faut dire que l'eau constitue indéniablement l'un des défis les plus importants de notre siècle ; cette ressource devient rare dans certaines zones de notre planète et représente un enjeu majeur de santé publique. Si les sujets en lien avec le réchauffement climatique traitent à juste titre des énergies lors des conférences internationales, la place de l'eau y est paradoxalement moins présente, reconnaissons-le, y compris dans le compromis final de la COP21. Pourtant, chaque être humain devrait pouvoir satisfaire ses besoins essentiels en eau, ce qui est loin d'être le cas. Sur la planète, près de 1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et plus de 2 milliards ne bénéficient pas d'un assainissement de base. Chaque année, plus de 2 millions de personnes meurent dans le de maladies liées à l'absence ou à la mauvaise qualité de l'eau. En France, grâce notamment à l'existence d'une politique volontaire, l'accès à l'eau et à l'assainissement est garanti au plus grand nombre, au plus grand nombre, mais seulement au plus grand nombre, car, hélas, tous ne bénéficient pas de ce droit fondamental. Entre 100 000 et 150 000 personnes, parmi les plus vulnérables et les plus démunis, en sont écartées, écartées, et l'on estime à près de 1 million les ménages ayant, certes, accès à l'eau, mais à un coût dont le niveau est jugé inabordable. Dès lors, comment ne pas saluer l'initiative des sept députés à l'origine de ce texte l'important travail de réflexion engagé par les lanceurs d'alerte que sont les associations et ONG regroupées au sein de la plateforme coordonnée par la fondation France Libertés et la Coalition Eau ? Je crois savoir que ce fut là le dernier, mais le plus beau des combats de Danielle Mitterrand. Force est de constater que ce droit à l'eau n'était pas encore formellement reconnu en France comme un véritable droit, bien qu'il bénéficiât d'une reconnaissance de principe dans plusieurs textes. Il y avait donc urgence sociale à faire de l'accès à l'eau un droit effectif pour tous. Dans cet objectif, la proposition de loi prévoit plusieurs mesures, dont la création et le financement d'une aide forfaitaire préventive pour l'eau en faveur des personnes en situation de précarité. C'est effectivement là, monsieur le rapporteur, qu'est le coeur du texte. En effet, les réponses apportées jusqu'à présent portaient, pour l'essentiel, sur le curatif, curatif, les CCAS ou les fonds de solidarité pour le logement, avec les limites que comportent de tels outils : procédures inégalitaires selon les départements et souvent considérées comme humiliantes ou stigmatisantes pour les ayants droit. De fait, il était difficile d'assurer une mise en oeuvre complète et équitable de ce droit. D'où la nécessité de ce volet préventif dans le présent texte, pour que le droit à l'eau soit un droit pour quel que soit son territoire de vie. Bref, il s'agit d'un dispositif de solidarité, qui devait être national, préventif et simple pour les bénéficiaires du RSA socle ou de la CMU complémentaire. Il était par ailleurs important de mobiliser les collectivités locales sur cette question éminemment sociale. Plusieurs dispositions complètent ainsi le code de la santé publique, afin d'obliger les collectivités territoriales et les EPCI à prendre les mesures nécessaires

les élus locaux n'ont pas attendu l'initiative de quelques députés hors sol pour organiser la solidarité sur leur territoire. Au contraire de la logique de ces dispositions, le suivi de ces questions par le CCAS, organisme local, permet d'accompagner les foyers fragilisés, et cette proximité garantit que l'aide offerte soit en adéquation réelle avec les besoins exprimés. Croyez-moi, cela sera toujours plus efficace qu'un dispositif complexe et bureaucratique le texte issu de la commission souffre d'un autre anachronisme : il a le côté « » de la France jacobine d'hier et de son hyper-réglementation.

Ainsi, mes chers collègues, je voterai contre ce texte, mais, dans une logique constructive, j'invite M. le rapporteur et M. le secrétaire d'État à prendre connaissance des propositions faites par le groupe de travail sur la simplification législative du droit de l'urbanisme, de la construction et des sols, où ils trouveront une inspiration pour le futur. De même, en consultant le texte de la proposition de résolution adoptée hier dans cet hémicycle sur l'initiative de notre collègue Rémy Pointereau, visant à améliorer la gestion de l'eau, ils trouveront des idées pour rendre l'eau moins chère et mieux distribuée, au service de tous.

cette proposition de loi repose sur des valeurs de solidarité et de générosité. On peut s'en féliciter, mais, en pleine campagne électorale, cela peut aussi sembler gratifiant pour ses auteurs Or le pragmatisme doit guider nos travaux et nous donner la faculté de nous abstraire de considérations dont l'unique vertu serait de flatter nos propres consciences tout en essayant de séduire les électeurs. Ce texte est la triste mais habituelle illustration de cette incapacité à résister aux propositions d'affichage dont les mesures sont à la fois inutiles et contre-productives. Elles sont d'abord

dans le cadre du Fonds de solidarité pour le logement, une ligne budgétaire a vocation à aider les familles en difficulté ; en 2010, 10 millions d'euros ont ainsi été consacrés à la prise en charge des impayés d'eau. N'oublions pas non plus la loi de notre excellent collègue François Brottes de 2013, qui prévoit une expérimentation sur cinq ans ; cinquante collectivités se sont portées volontaires. Aussi, ne brûlons pas les étapes, expérimentons !

Aussi, mes chers collègues, je ne me laisserai pas séduire par ce texte, je voterai contre cette proposition de loi, qui me semble inutile, puisque les outils existent déjà, ... Mais non ! ... et parce que je souhaite que l'on continue de faire confiance aux élus locaux.

pourra largement être remise en question. Ensuite, elle pourrait bouleverser l'équilibre qui résulte des dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code général des collectivités territoriales sur le service public de l'eau et de l'assainissement et de la jurisprudence y afférent. les dispositions précitées prévoient que les communes arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution, c'est-à-dire les zones dans lesquelles l'obligation de desserte s'applique. Par voie de conséquence, si une construction ne figure pas dans une telle zone desservie par le réseau distribution, la commune n'a pas d'obligation de raccordement. Tel est le sens donné à ces dispositions par le Conseil d'État, qui a considéré qu'une collectivité territoriale n'a pas l'obligation

par la volonté de supprimer l'article 1. Je n'avais pas compris que la majorité sénatoriale souhaitait détricoter le bilan international de l'ancien président ... Il se trouve en outre

Cette crainte n'est pas fondée, car les compétences des collectivités territoriales en matière d'assainissement collectif et non collectif ne sont pas remises en cause. Les collectivités auront toujours la responsabilité de l'établissement des zones d'assainissement non collectif en tenant compte de l'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique et des coûts que représente une installation collective, comme cela est prévu dans le code général des collectivités territoriales. Le Gouvernement est donc défavorable défavorable à la suppression de cet article, qui permet notamment de définir le droit d'accès à l'eau et de mettre en cohérence les différents codes traitant de ce sujet. La parole

que vous n'avez vraiment pas envie d'appliquer ce droit fondamental à l'eau pour tous. Remarquez, au moins, vous êtes cohérents

L'article 1 dispose simplement que le droit à l'eau potable et à l'assainissement comprend le droit, pour chaque personne physique dans des conditions compatibles avec ses ressources, de disposer chaque jour d'une quantité suffisante d'eau potable pour répondre à ses besoins élémentaires ; d'accéder aux équipements lui permettant d'assurer son hygiène, son intimité et sa dignité. L'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics concourent à la mise en oeuvre du droit à l'eau potable et à l'assainissement.

En effet, si nombre de nos concitoyens n'ont pas accès à l'eau potable et à l'assainissement, nous le devons d'abord à un manque structurel de places d'hébergement d'urgence et, plus généralement, à une crise du logement, qui se traduit par un déficit chronique de constructions de logements, en premier lieu de logements sociaux. sociaux. Ainsi, en décembre 2013, 43 % des sans domicile fixe qui ont composé le 115 n'ont pas obtenu de place à Paris,

les réseaux d'eau potable notamment, avant de penser à construire des installations dont on ignore si elles seront finalement utilisées.

Les problèmes auxquels le texte veut apporter une solution se posent à l'évidence, et pour l'essentiel, dans les métropoles, métropoles dont une récente étude de France Stratégie

aujourd'hui ? Est-ce que vous croyez que vous allez résoudre le problème des SDF d'ici à deux ou trois semaines ? Non !

Si l'on peut être favorable à l'existence d'un traitement curatif des difficultés que peuvent éprouver nos concitoyens pour avoir accès à l'eau et à l'assainissement, à travers la prise en charge des impayés par les centres communaux d'action sociale- on le fait régulièrement dans nos communes pour régler un certain nombre de problèmes -ou les fonds de solidarité pour le logement, qui ont été institués par la loi de 1990 et qui relèvent des conseils généraux depuis 2004, l'introduction de deux mécanismes d'aide préventive avec l'aide préventive pour l'eau et la création d'une allocation forfaitaire d'eau pour les ménages les plus pauvres participe, une fois de plus, à un long processus de déresponsabilisation de nos concitoyens. Cette déresponsabilisation est puisqu'il va falloir anticiper des situations d'impayés consécutives, soit à un prix de l'eau trop élevé- comme le prévoit le mécanisme d'allocation forfaitaire d'eau -, soit à des dépenses d'eau trop importantes au regard des ressources des ménages- comme le prévoit l'aide préventive pour l'eau mentionnée à l'article 3.

le Sénat avait adopté à l'unanimité, en décembre 2011, un article 16 C nouveau dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2011, aux termes duquel l'aide préventive en matière d'accès à l'eau était financée par une contribution de 1 % sur les recettes des services d'eau et d'assainissement. Répondant à la demande émanant de l'opposition, mais aussi de nombreux députés de la majorité de l'époque qui réclamaient la création d'un volet préventif pour l'aide à l'eau, la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet déclarait, le 1 décembre 2010, à l'Assemblée nationale : « Je le redis ici solennellement : nous sommes déterminés à ajouter un volet préventif au volet curatif [ ...] construit sur un schéma du type allocation APL. » Saisi en février 2011 par les ministres Nathalie Kosciusko-Morizet et Roselyne Bachelot, le Conseil général de l'environnement et du développement durable publia, quelques mois plus tard, une étude intitulée.

est le plus essentiel, la coupure d'eau rendant les conditions de vie totalement inacceptables. [ ...] C'est pourquoi il est indispensable de mettre en place une véritable action préventive.

la commission a émis un avis favorable

pour l'accès à l'eau ». Or les fonds de solidarité pour le logement départementaux peuvent déjà aider les personnes physiques qui se trouvent « dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau,

le produit de cette taxe est affecté au régime vieillesse de base des non-salariés agricoles. Compte tenu du déficit structurel annuel de 300 millions d'euros de ce régime et de son passif cumulé- plus de 3 milliards d'euros de dettes financées par emprunt

Pourtant, dans ces départements, il y a aussi des gens qui ont besoin d'avoir accès à l'eau. Lorsque le volet « eau » des FSL est abondé, les montants disponibles sont parfois insuffisants. Cela figure dans le rapport du Conseil

La séance est suspendue. La séance est reprise. Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat qu'il a été saisi le 22 février, en application de l'article 54 de la Constitution, par plus de soixante députés, de l'accord économique et commercial global, ou AEGG, entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part. Le texte de la saisine est disponible au bureau de la distribution. Acte est donné de cette communication.

le groupe de l'UDI-UC a souhaité inscrire dans la « niche » lui étant réservée un temps d'échange et de débat sur la problématique des déserts médicaux et la présence des professions paramédicales. Le constat de l'existence de déserts médicaux n'est pas nouveau.

Dans mon département, la Haute-Loire, si l'on cherche un spécialiste sans dépassement d'honoraires, l'accès aux soins est des plus difficiles. La Haute-Loire n'est toutefois pas la plus démunie face à la désertification médicale. D'autres départements doivent faire face à des situations bien plus préoccupantes. Malheureusement, ne pas répondre à la désertification médicale, c'est prendre le risque de voir celle-ci s'étendre à d'autres professions de santé, ce qui est déjà le cas dans certains départements. L'accès équitable aux soins est devenu l'une des préoccupations majeures de nos concitoyens. De nombreux dispositifs ont déjà vu le jour pour tenter d'y remédier depuis une quinzaine d'années. à la loi HPST en 2009 ou à la loi Santé en 2016. À ce sujet, mes chers collègues, je tiens à souligner que de nombreux décrets d'application ne sont pas pris, rendant ces textes, pourtant très novateurs, inapplicables. La face cachée des déserts médicaux ne serait-elle pas due aussi à l'inapplication de la loi ? De ces différentes lois, il convient de distinguer les mesures incitatives et ponctuelles, visant à rendre plus attractives les zones sous-médicalisées, des mesures structurelles, qui portent sur l'organisation générale de l'offre de soins. Des dispositifs incitatifs ciblés ont été proposés, comme les exonérations fiscales et sociales financées par l'État pour l'installation dans certaines zones- ZRR ou ZRU - ; la loi du 23 février 2005 prévoit également une exonération d'impôt sur le revenu au titre de la participation à la permanence des soins. Les professionnels de santé bénéficient également d'incitations à l'installation en zones sous-dotées financées par l'assurance maladie- le contrat d'engagement de service public -ainsi que de nombreuses aides financées par les collectivités territoriales qui peuvent prendre des formes diverses : la prise en charge de tout ou partie des frais d'investissement ou de fonctionnement liés à l'activité de soins, la mise à disposition de locaux destinés à cette activité, la mise à disposition d'un logement et bien d'autres. En contrepartie de ces aides, leurs bénéficiaires doivent s'engager à conserver leur activité dans la même zone pendant trois ans. Leur engagement est matérialisé par une convention tripartite passée entre la collectivité territoriale, l'assurance maladie et le professionnel de santé. La nouvelle convention médicale de 2016 propose ainsi la mise en place de contrats d'installation, de contrats de transition, de contrats de stabilisation et de coordination. L'empilement de l'ensemble de ces dispositifs se traduit parfois par une absence totale de lisibilité et par une impossibilité d'évaluation des coûts. La Cour des comptes elle-même n'y est pas parvenue. Notre système de santé est confronté à un double défi, démographique et économique. À côté de ces mesures dites « incitatives » existent les mesures dites « structurelles », comme la nouvelle organisation de la permanence des soins, qui permet une prise en charge la nuit, les week-ends et les jours fériés. Toutefois, cette permanence des soins n'est pas, en tant que telle, une solution à la difficulté croissante dans certaines zones pour consulter un médecin dans des conditions raisonnables de distance et de délais. Je tiens aussi à évoquer le soutien au développement des maisons et pôles de santé. Les maisons et pôles de santé pluriprofessionnels semblent une réponse possible de réorganisation de la médecine de premier recours. Les médecins libéraux montrent depuis longtemps une préférence pour l'exercice regroupé, qui est désormais devenu le mode d'exercice majoritaire. Ces maisons de santé réunissent dans des locaux communs plusieurs médecins généralistes, infirmiers et d'autres professionnels de santé exerçant à temps plein ou à temps partiel : médecins spécialistes, dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, podologues, diététiciens, psychologues, orthophonistes et autres Néanmoins, les maisons de santé contribuent d'une certaine manière à accélérer le processus de concentration géographique des professionnels de santé. Ces structures peuvent aider à maintenir la présence de ceux-ci dans les zones en voie de fragilisation, mais ne peuvent pas répondre aux besoins des zones déjà désertées. Lutter contre les déserts médicaux, mes chers collègues, c'est avant tout lutter contre la désertification rurale, en rendant la ruralité attractive. Ce n'est pas Alain Bertrand qui me démentira Nous devons renforcer l'attractivité des territoires affectés par l'absence d'une offre de soins cohérente, critère déterminant pour choisir de s'installer ou non sur un territoire. Sans politique d'aménagement du territoire ambitieuse, toute mesure incitative est vouée à l'échec.

du nombre de médecins par habitant, nous reviendrons aux chiffres de 1985, soit 283 médecins pour 100 000 habitants. Les solutions déjà proposées visant à interrompre la désertification médicale se sont révélées pour l'instant inefficaces, voire contre-productives.

Pour lutter contre le manque de médecins, des améliorations sont pourtant possibles, notamment grâce au partage de l'activité médicale entre praticiens et professions paramédicales. La légitimité de ce transfert est venue de la compétence que ces acteurs ont acquise, sans en avoir obtenu la reconnaissance. Afin d'encadrer et de développer ces pratiques, tout en donnant à leurs acteurs la légitimité nécessaire, la loi du 26 janvier 2016 a ouvert la possibilité à certaines formes de délégation, entendues comme la réalisation d'activités entrant dans le champ d'activité du médecin par un professionnel paramédical non-médecin. Ces délégations doivent être précisément définies par décret en Conseil d'État et peuvent concerner les activités d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage les actes d'évaluation et de conclusion clinique, les actes techniques et les actes de surveillance clinique et paraclinique, ainsi que les prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire, les prescriptions d'examens complémentaires et les renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales. Les professions paramédicales concernées sont nombreuses. Les conditions et règles de ces nouvelles pratiques, ainsi que les diplômes nécessaires pour leur exercice, délivrés par des universités préalablement habilitées à cet effet, doivent également être fixées par décret. L'accélération des transferts de compétences permettra de mieux réguler les files d'attente, de faire partiellement face à la diminution annoncée de la démographie médicale. Ce transfert permet également d'optimiser le système de soins, d'éviter la mise en place d'organisations parallèles, sources de conflits et de baisse de la qualité des soins, et d'apporter une légitime reconnaissance à certains professionnels paramédicaux. En matière d'optique correctrice, le transfert de certains actes vers les orthoptistes permet déjà de diminuer les délais d'attente. Pharmaciens et infirmiers s'établissent là où existent des besoins, ce qui n'est pas le cas des médecins. Nous devons nous servir de ce maillage territorial pour pallier le manque de médecins. Promouvoir l'exercice pluriprofessionnel coordonné est la piste à privilégier. Les professionnels pourraient se mettre d'accord sur les conditions de renouvellement d'ordonnances par les pharmaciens ou sur les interventions plus importantes des infirmières en ce qui concerne le suivi des patients à domicile. En France, les formations de santé sont de très haute qualité, mais des améliorations sont nécessaires pour permettre aux futurs professionnels de santé d'acquérir des fondamentaux partagés pour une meilleure prise en charge du patient. Il me semble essentiel, mes chers collègues, de développer chez les étudiants une culture du travail en commun entre les secteurs médical et paramédical, en organisant des rendez-vous pluridisciplinaires autour de cas cliniques. Cette démarche pourra rapprocher l'université des instituts de formation paramédicale. Dès cette année, les diplômés paramédicaux pourront avoir accès aux deuxième et troisième années de médecine, en suivant les mêmes procédures que l'ensemble des étudiants. Un kinésithérapeute pourrait ainsi, « sur la base d'un projet solide ou sur dossiers », suivre des études de médecine pour devenir médecin rééducateur. Le monde paramédical emploie plus de 1 million de personnes, et la liste des recruteurs potentiels est longue. Sans être médecins, les professionnels paramédicaux dépistent des problèmes de santé, contribuent aux soins et à l'amélioration des conditions de vie du patient. Les compétences s'étoffent, notamment pour les infirmiers, qui se voient confier de nouvelles tâches, comme le suivi du traitement de maladies chroniques. Le rôle des paramédicaux dans la prise en charge de la dépendance est moins connu. Pourtant, ces professionnels jouent un rôle important dans la prise en charge pluridisciplinaire des personnes âgées dépendantes.

face à la dégradation de la médecine libérale et à la désertification médicale, le constat est qu'à ce jour aucune réforme ne parvient à endiguer les problématiques touchant notre système de santé. Des améliorations sont possibles, notamment grâce au partage de l'activité médicale entre praticiens et professions paramédicales, voire au développement du travail collaboratif. La parole

débat s'inscrit dans la continuité de celui qui s'est tenu dans cet hémicycle le 7 avril 2016 sur l'offre de soins dans les territoires ruraux

les premiers étudiants concernés par le fameux instauré en 1971 prennent leur retraite en ce moment, ce qui explique, pour une large part, la situation actuelle. Le relèvement du en 1999 fut trop tardif et explique le creux que nous connaissons. Ensuite, la formation des médecins a évolué, en particulier celle du généraliste, qui n'est plus initié aux gestes de la médecine polyvalente : petite chirurgie, gynécologie, pédiatrie, ORL,

Face à cette impasse structurelle, les réformes à engager sur la sélection des jeunes médecins, hommes et femmes, sur leur formation, sur le lieu de leurs premières expériences professionnelles, voire, si l'on ose, sur leur liberté d'installation, sont colossales promettent d'intenses batailles politiques et parlementaires. En tout état de cause, elles ne produiront de toute façon pas d'effets avant une décennie ou deux. Pour apporter une réponse conjoncturelle à ce problème, les deux derniers gouvernements ont créé et développé des maisons pluridisciplinaires de santé, dont le nombre devrait approcher le millier à la fin de l'année en cours. C'est, nous le pensons, une bonne méthode pour pallier une offre de soins insuffisante et inciter les médecins à s'installer en zone rurale. Certains envisagent même, dans la mesure du possible, de développer l'itinérance de ces maisons de santé, afin qu'elles puissent se déplacer au plus près des patients. Cependant, ce dispositif est loin de régler tous les problèmes, au regard du nombre de personnes aujourd'hui privées de médecins. Ces réflexions nous conduisent au débat du jour : les professions paramédicales peuvent-elles jouer un rôle pour combler une partie de cette absence d'offre de soins ? Sur le papier, la chose paraît tout à fait raisonnable. Nombre d'actes médicaux sont répétitifs et pourraient être effectués par des paramédicaux ayant reçu une formation initiale ou complémentaire adaptée.

gynécologique ou contraceptif des femmes. Il faut cependant faire preuve de prudence. En effet, si certains soins peuvent être délégués, la responsabilité de ces actes incombera toujours au médecin. On peut tout de même imaginer une évolution des pratiques dans un certain nombre de cas. Ainsi, certaines professions paramédicales pourraient tenir une place plus importante dans la coordination des soins, ainsi que le dépistage et le suivi de traitements au long cours. Les infirmiers, par exemple, pourraient se voir accorder un rôle accru dans le suivi des maladies chroniques. De la même manière, dans le cadre de protocoles élaborés avec un médecin, ils pourraient assurer un suivi plus fin des patients et être en mesure, par exemple, de renouveler les ordonnances. suivi devra néanmoins être encadré par des visites régulières chez le praticien. La délivrance de certificats d'aptitude, notamment sportive, pourrait aussi leur incomber.

de soi -, elle pourrait être renforcée par la présence de paramédicaux aux côtés du patient lors de la consultation virtuelle avec le médecin. D'autres pistes intéressantes concernant les ophtalmologistes, les orthoptistes, les oculistes ont également été imaginées et seraient bien utiles dans certaines régions. Pour conclure, je souhaite dire qu'il n'est pas interdit d'être pragmatique et réaliste pour faire face à la situation catastrophique de la répartition de l'offre de soins sur le territoire. Les paramédicaux peuvent, dans une certaine mesure, combler le manque de médecins généralistes. Mais soyons très clairs, si des solutions d'appoint peuvent être trouvées rapidement,

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui sur l'initiative de nos collègues

Nous attendons les résultats de leurs travaux avec beaucoup d'intérêt. En tant qu'élus locaux et nationaux, nous sommes confrontés quotidiennement aux effets de la désertification médicale et à l'inquiétude de nos concitoyens face au départ à la retraite du médecin du village qui ne comptait pas ses heures et ses jours au chevet de ses patients. Sera-t-il même remplacé ? De plus, on constate une interdépendance entre les professionnels de santé dans les zones sous-dotées. Lorsque le médecin généraliste disparaît du terrain, ce sont les professionnels paramédicaux qui suivent. Telle est la réalité. réalité. Le pharmacien est souvent le dernier rempart auprès des citoyens en tant que personnel de santé, mais, à moyen terme, il finit aussi par partir. La France compte actuellement 220 000 médecins, soit deux fois plus qu'en 1980.

devenir un désert médical en médecine générale, contre seulement 180 médecins pour 100 000 habitants dans l'Eure. Durant de nombreuses années, nous n'avons pas anticipé le changement des attentes des médecins concernant l'évolution de leurs pratiques professionnelles.

ont désormais besoin de coopération médicale avec d'autres professionnels de santé afin de répondre toujours mieux aux attentes des patients. La fin du modèle du médecin omniscient, exerçant seul, La demande de dialogue et d'échanges est dorénavant très forte chez les médecins, tant avec les acteurs du monde libéral qu'avec ceux du monde hospitalier. Depuis 2012, le Gouvernement a pris en compte ces évolutions et mené une politique volontariste de lutte contre les déserts médicaux. Je veux rappeler les dispositifs mis en place pour les nouvelles générations de médecins,

Pour lutter contre les déserts médicaux, il est primordial d'agir sur la formation des médecins. Il faut ainsi augmenter le nombre de maîtres de stages universitaires recrutés parmi les professionnels de santé de terrain, tant en milieu rural qu'en milieu urbain et dans les banlieues. mettre en place des contrats d'engagement de service public. Des bourses de 1 200 euros bruts par mois devraient être versées aux étudiants volontaires décidant de s'installer dans une région manquant de médecins. À ce jour, 1 800 jeunes médecins ont souscrit un tel contrat et s'installeront bientôt dans des territoires sous-dotés. Par ailleurs, 650 médecins ont signé un contrat de praticien territorial de médecine générale. En contrepartie de leur installation, ils bénéficient de nouvelles garanties, en particulier d'une protection sociale améliorée.

Après avoir évoqué les outils de lutte contre la désertification médicale, j'aborderai plus spécifiquement maintenant le rôle des professions paramédicales dans la lutte contre les déserts médicaux. Ce rôle, cela a rôle, cela a été dit, est éminent dans le cadre des maisons pluriprofessionnelles de santé. Je suis convaincue, en tant que professionnelle de santé, de l'importance des coopérations médicales interprofessionnelles. Il est nécessaire de lutter contre les corporatismes qui s'expriment encore fortement, osons le dire, mais également de valoriser la qualité des métiers et leurs évolutions possibles. Je n'ignore pas qu'un certain nombre de malaises s'expriment au sein des professions paramédicales chez les infirmiers et les aides-soignants, mais aussi chez les étudiants orthophonistes, qui ont récemment réclamé certes des revalorisations salariales, mais surtout de meilleures conditions de travail et une reconnaissance de leur activité.

cette qualification d'infirmier clinicien étant la porte ouverte aux coopérations interprofessionnelles. Par ailleurs, les conditions de prise en charge de nos concitoyens, médecine et en chirurgie ambulatoire par exemple, vont entraîner tant pour les médecins que pour les personnels paramédicaux des coopérations beaucoup plus abouties qu'aujourd'hui entre l'hôpital et la ville. Le parcours de santé de nos concitoyens Ainsi, les auxiliaires médicaux formés à assumer des pratiques avancées doivent exercer dans des équipes de soins en lien avec le médecin traitant afin d'améliorer la réponse aux besoins des patients chroniques.

prescriptions d'examens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales. Dans ce cadre, les sages-femmes, profession médicale rappelons-le, ont vu leurs responsabilités reconnues dans le suivi des grossesses normales. Les professionnels paramédicaux dans leur ensemble se plaignent des difficultés de leurs conditions de travail. Pour répondre à ce malaise, le Gouvernement a présenté en décembre 2016 une stratégie nationale d'amélioration de la qualité de vie au travail devant permettre la définition de bonnes conditions de vie au travail et la détection des risques psychosociaux. Avant de terminer mon propos, il me semble fondamental d'intégrer dans nos réflexions les innovations radicales dont va bénéficier notre système de santé : les nanotechnologies, les biotechnologies, les capacités informatiques, les sciences cognitives. Les avancées réalisées en télésanté, en intelligence artificielle et en génétique vont modifier considérablement la médecine de demain, ainsi que son enseignement. Au-delà de la connaissance des progrès de la science et de leur déclinaison dans la pratique, par exemple l'apprentissage de l'utilisation d'un robot chirurgical, les sciences humaines doivent occuper une large part dans tous les métiers qui concernent la santé. j'évoquerai les visio-consultations. On peut imaginer qu'à un horizon prochain, dans une dizaine d'années sans doute, elles constituent la principale porte d'entrée des parcours de soins.

Les professionnels paramédicaux, dont je veux ici saluer une nouvelle fois l'engagement total de proximité, au quotidien, auprès de nos concitoyens, expriment parfois un certain mécontentement : leur reconnaissance statutaire n'est pas totale, elle ne va pas assez vite, leurs conditions de travail sont difficiles. J'ai tout à fait conscience de tout cela, mais je souhaite que ces professionnels fassent des propositions aux candidats à l'élection présidentielle. Nous avons reçu les uns et les autres les propositions des masseurs-kinésithérapeutes,

les professions paramédicales pourraient jouer dans la lutte contre les déserts médicaux fait écho à un rapport d'information sur la coopération entre professionnels de santé que j'ai présenté, avec notre collègue Catherine Génisson, au nom de la commission des affaires sociales en 2014. Cette question fait également écho à un débat qui s'est tenu lors de la discussion de la loi de modernisation de notre système de santé, dont l'une des mesures vise à créer un exercice en pratique avancée pour les professions paramédicales. Permettez-moi de revenir rapidement sur ce qui existe déjà en matière de coopération entre professionnels de santé et pratique avancée pour les professions paramédicales. Dès le début des années 2000, de nombreux travaux et rapports, je pense notamment à ceux du professeur Yvon Berland, ont pointé le retard de la France en matière de ce que l'on désignait alors sous le nom de « transferts de tâches », alors même qu'il existait une réelle volonté de certains acteurs médicaux et paramédicaux de l'organiser. La loi a ensuite prévu la mise en oeuvre de protocoles expérimentaux de coopération entre professionnels. Je fais référence à l'article 51 de la loi HPST de 2009. Cette mesure a contribué à faire évoluer les esprits. Les enseignements tirés de la mise en oeuvre de ces protocoles montrent qu'une évolution structurelle des métiers de la santé est souhaitable, à la fois pour une meilleure efficacité pour les patients et pour une plus grande satisfaction des professionnels de santé. Force est de constater que la répartition des compétences entre les différentes professions de santé est trop rigide. Elle freine ainsi la continuité entre les compétences et les niveaux de responsabilité reconnus aux médecins, d'une part, et aux autres professions de santé, d'autre part. Cette situation est fortement préjudiciable à l'attractivité des métiers de santé : tandis que les jeunes générations de médecins aspirent à organiser différemment le temps temps médical, les autres professions médicales et paramédicales réclament davantage de reconnaissance, d'autonomie et de possibilités d'évolution de carrière. Nous avions clairement identifié, lors de l'élaboration du rapport d'information de 2014, les effets néfastes qu'une telle situation provoque, à savoir une frustration professionnelle, d'une part, et une déperdition de compétences, d'autre part. Par ailleurs, nous avions souligné qu'un maillon de la chaîne des compétences en matière de soins manquait, celui des qualifications intermédiaires. Entre les médecins formés de neuf à dix ans après le baccalauréat et les auxiliaires médicaux formés de deux à trois ans, parmi les professions paramédicales, il n'existe que très peu de métiers de santé sanctionnés par un niveau d'études de cinq ans. Il existe des infirmiers spécialisés en anesthésie et en chirurgie, dont le diplôme d'État est équivalent à un grade de niveau master, mais peu de professions intermédiaires. Or les enjeux attachés à une évolution de cette structuration sont d'importance. Cependant, contrairement à une idée reçue, les protocoles de coopération entre professionnels de santé n'ont pas comme objectif premier de remédier aux difficultés posées par la démographie médicale. Si une nouvelle répartition des compétences entre médecins et autres professionnels médicaux ou paramédicaux peut effectivement aboutir à dégager du temps médical, elle ne saurait compenser qu'à la marge l'absence de professionnels dans les zones sous-denses. Par ailleurs, il serait erroné de réduire la question des coopérations à un débat entre médecins d'un côté et autres professionnels de santé de l'autre. La question de la répartition des actes se pose pour l'ensemble des professions de santé, quel que soit le niveau de formation initial requis. Plus récemment, comme je le rappelais au début de mon intervention, l'article 119 de la loi de modernisation de notre système de santé a créé un exercice en pratique avancée pour les professions paramédicales. Nous avions approuvé cette mesure puisqu'elle était la traduction législative de la sixième proposition formulée dans le rapport d'information de la commission des affaires sociales. En ma qualité de rapporteur, j'avais cependant regretté que cet article se limite à un toilettage du statut de certaines professions paramédicales alors qu'il aurait pu être l'occasion d'une remise à plat des métiers socles. En l'état actuel, pour chaque auxiliaire médical, des mesures réglementaires doivent définir les domaines d'intervention en pratique avancée, les activités pouvant être accomplies dans chacun de ces domaines d'intervention et les types d'actes pouvant être réalisés. Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous informer de l'état d'avancement de ces mesures ? La mise en oeuvre effective de l'article 119 est en effet essentielle puisqu'il s'agit aussi d'améliorer la qualité des soins en confiant davantage de compétences aux professionnels paramédicaux que sont notamment les infirmiers. Avec le développement des affections chroniques, notamment les cancers et les maladies cardio-vasculaires, et la progression des pathologies liées au vieillissement, les besoins des malades évoluent vers une prise en charge plus globale et de plus grande proximité. À Lille, par exemple, il existe un protocole de soins de suite en cancérologie reposant sur les infirmières libérales. Il faut donc développer ces coopérations dont l'apport est double. D'une part, elles tendent à améliorer la qualité des soins en offrant une prise en charge plus adaptée aux besoins des patients, en apportant le plus souvent des innovations en matière de prise en charge, en impliquant par exemple la création de nouveaux actes ou de nouvelles formes de prise en charge. D'autre part, elles offrent à tous les professionnels une perspective d'évolution de leur rôle en matière de soins, ainsi qu'un enrichissement de leurs tâches susceptible de renforcer leur motivation et leurs perspectives de carrière. Pour conclure, j'indique qu'il est nécessaire de développer le rôle des professions paramédicales dans un système de santé qui doit s'adapter pour répondre aux nouveaux enjeux de ce début du XXI XXI siècle que sont les transitions démographique, épidémiologique et technologique, comme l'a dit Catherine Génisson. Il importe aussi d'encourager davantage, d'une manière forte et volontaire, l'e-santé, dont le développement dans les pays voisins de la France montre qu'elle est efficace, complémentaire de l'humain. Elle permettra rapidement de rationaliser l'offre de soins sur nos territoires puisque certains pensent, et l'ont écrit, que 80 % des diagnostics pourraient être faits par celle-ci. La

la lutte contre les déserts médicaux, sujet que nous n'avons pas l'habitude d'aborder sous cet angle. En effet, nous parlons davantage du manque de médecins, de sages-femmes, de dentistes ou de pharmaciens, c'est-à-dire des professions médicales, dans les territoires et des mesures incitatives ou contraignantes pour combattre les déserts médicaux. Je remercie donc le groupe de l'UDI-UC d'ouvrir ce débat aux professions paramédicales que je connais bien, étant moi-même orthophoniste. En France, selon les données de la DREES, au 1janvier 2015, plus de 1 million de personnes exercent une profession paramédicale, soit près de 640 000 infirmiers, plus de 400 000 aides-soignants et 154 500 professionnels de la rééducation. Les professionnels du secteur accompagnent, préparent, soignent, appareillent et rééduquent les patients selon leur spécialité : la diététique, la puériculture, les soins infirmiers, la kinésithérapie, l'orthophonie, etc. Les professionnels du secteur paramédical sont majoritairement salariés, du secteur public, privé ou associatif. Ils travaillent dans les hôpitaux et les cliniques, les centres médico-sociaux, les centres de santé, les maisons de retraite, les cabinets médicaux, les centres d'imagerie médicale, etc. Chaque année, certains secteurs comme la gériatrie ou la psychiatrie et certaines régions, rurales ou urbaines, je pense notamment à l'Ile-de-France, peinent à recruter et à fidéliser les professionnels du secteur.

comme celui de responsable de service de soins à domicile. Pour faire face à ces nouveaux besoins dans les territoires, il est indispensable de revoir la formation des professions paramédicales en donnant aux facultés les moyens de formation nécessaires pour accueillir davantage d'étudiants. Or de Or de nombreuses écoles d'infirmiers ont, au contraire, été fermées par les pouvoirs publics. D'un côté, les besoins augmentent, de l'autre, les capacités d'accueil se réduisent pour les formations des paramédicaux. À cela s'ajoute l'absence de reconnaissance de la formation paramédicale à son juste niveau. Actuellement, la plupart des professions paramédicales nécessitent un cursus de trois à cinq ans après le bac qui ne fait pas l'objet d'une transposition dans le cadre universitaire LMD, ce qui est profondément injuste. Ainsi, les cursus paramédicaux de manipulateur en électroradiologie et de pédicure-podologue, le DST en imagerie médicale n'ont toujours pas été

Un étudiant qui décide d'exercer son métier à l'issue de ses études de kinésithérapie ne pourra revendiquer qu'un master 1. Pour être reconnu master 2, il devra poursuivre des études à l'issue de sa formation en institut de formation en masso-kinésithérapie. Ce problème de reconnaissance des qualifications touche également les orthophonistes, dont la formation a été reconnue bac+5 au grade master 2 depuis 2013 sans que cette reconnaissance se soit accompagnée d'une revalorisation salariale. Les orthophonistes restent rémunérés, dans les établissements publics, sur la base d'un niveau bac+2, entre 1 200 et 1 300 euros nets, soit à peine plus que le SMIC, en début de carrière. Ces mêmes professionnels sont soumis au, alors qu'on manque partout cruellement d'orthophonistes. Aux difficultés de formation et de reconnaissance des qualifications que connaissent les professions paramédicales s'ajoutent des conditions de travail souvent tendues et difficiles. Ces professions subissent les réductions budgétaires imposées par l'État dans le domaine de la santé. Cette précarité touche aujourd'hui majoritairement des femmes, puisqu'une quinzaine de métiers du secteur paramédical sont exercés à plus de 80 % par des femmes. Mal vécue à juste titre, cette précarité peut être à l'origine d'une reconversion. C'est ainsi que, en 2011, près de 10 % des infirmières ont quitté l'hôpital public et changé de métier. On le constate, il s'agit donc non seulement de revoir les formations, mais de revaloriser toutes ces professions paramédicales en leur accordant un statut correspondant aux missions accomplies avec des salaires nettement réévalués,

et citoyen pensent que, pour s'assurer de la présence des professionnels paramédicaux partout avec un véritable maillage territorial, il faut instaurer un service public des soins de premiers recours. Ceux-ci doivent pouvoir s'exercer en lien avec des centres de santé- je parle bien de « centres de santé », non de « maisons de santé ». C'est pourquoi nous proposons que chaque bassin de vie soit pourvu d'un centre de santé regroupant des professionnels médicaux et des professionnels paramédicaux, d'où l'importance d'une action volontariste de l'État en termes de moyens. À la différence des maisons de santé, les centres de santé permettent un accès à toutes et tous avec une prise en charge à 100 % par la sécurité sociale grâce à la pratique du tiers payant et au respect des conventions en secteur 1. Nous sommes convaincus que ces structures répondent non seulement aux besoins des populations sur les territoires qui aspirent à pouvoir faire appel à des professionnels paramédicaux, également aux aspirations des professionnels paramédicaux qui souhaitent travailler en équipe. Cette pratique facilite coopération et coordination pluriprofessionnelle, ce qui simplifie le suivi global du patient et permet de développer des actions de prévention et d'éducation. Un autre argument qui plaide en faveur des centres de santé, c'est, comme pour les professions médicales, la volonté des jeunes praticiens de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Je conclurai mon propos en soulignant que les professionnels de santé ont tendance à s'installer, à juste titre, dans le périmètre de structures hospitalières.

conséquent bien celui de mener une autre politique de santé que celle qui est conduite depuis des décennies et, fâcheusement, depuis la loi Bachelot amplifiée par la loi Touraine que le Sénat comme l'Assemblée nationale ont, hélas, votée à l'exception de mon groupe, faut-il le rappeler La colère des personnels de santé est forte, et ils seront nombreux le 7 mars prochain à Paris pour le dire. Je serai à leurs côtés, ainsi que l'ensemble de mon groupe,

tant à l'hôpital qu'en secteur libéral. Toutefois, dans les zones périurbaines, on peut avoir rapidement accès, grâce aux transports, à un territoire mieux équipé en matière de santé, comme tandis que, dans les territoires hyper-ruraux, c'est beaucoup plus compliqué à cause de l'éloignement. Il faut donc trouver un moyen de remédier sur place à la pénurie médicale.

permet la mise en place, sur l'initiative des professionnels, à titre dérogatoire et expérimental, de transferts d'actes ou d'activités de soins. Les personnels paramédicaux engagés dans l'expérimentation sont formés

sur l'ensemble du territoire. Eh oui ! Autre problème : si, dans la hiérarchie des normes, la loi est supérieure au règlement, nombre de décrets, comme celui de 2004 relatif aux infirmiers diplômés d'État, n'ont pas été « toilettés » pour intégrer la possibilité expérimentale et dérogatoire prévue dans la loi Hôpital. En conséquence, les blocages persistent. Par exemple, les piqûres par injection sont réservées aux infirmiers diplômés d'État et interdites aux aides-soignantes, alors que celles-ci pourraient réaliser sans danger des injections sous-cutanées et intramusculaires. Parallèlement, il existe des avancées dans les délégations de compétences. Ainsi, dans certaines cliniques ou certains centres hospitaliers, des actes très techniques, comme les biopsies en cancérologie, sont réalisés par des infirmiers diplômés d'État. En imagerie, des actes d'échographie peuvent être accomplis par des manipulateurs radio dans un cadre très précis. Sur le terrain, les orthoptistes effectuent de nombreuses tâches réservées autrefois aux seuls ophtalmologistes. Les possibilités de délégations aux personnels paramédicaux sont donc multiples. Malheureusement, les choses évoluent lentement. Il faut en moyenne quatre ans pour obtenir une expérimentation, ce qui décourage les professionnels. Quels sont les

Il faut avant tout dépasser les visions « défensistes » et corporatistes de chacun des métiers. On peut évoquer notamment deux pistes. Une première piste consisterait à améliorer les procédures existantes prévues à l'article 51 de la loi Hôpital : accélération du délai d'approbation des protocoles, généralisation à l'ensemble du territoire de tout protocole validé par la Haute Autorité de santé, ou encore toilettage des décrets relatifs à chaque profession paramédicale. seconde piste est la création de nouveaux métiers de la santé qui pourraient prendre en charge de façon pérenne des tâches dévolues autrefois aux médecins et encadrées strictement. Je pense notamment au droit de prescription pour le renouvellement ordinaire de certains traitements qui, là encore, permettrait d'alléger la tâche des médecins et de leur redonner du temps. Quoi qu'il en soit, le domaine de la délégation ne peut être pensé que globalement, c'est-à-dire en organisant intelligemment une cascade de délégations.

Les blocages sont essentiellement liés à des peurs inhérentes aux compétences, à des réflexes corporatistes et quelquefois à du mépris. Ce sont des professions particulières À la cascade de méfiance et de mépris, il faut substituer une cascade vertueuse de délégations confiantes et constructives.

je veux bien sûr féliciter Olivier Cigolotti, qui a proposé au groupe de l'UDI-UC, auquel j'ai l'honneur d'appartenir, l'organisation de ce débat, qui est particulièrement pertinent quand on sait combien est essentielle la question de la désertification médicale. désertification médicale. Je regrette à cet égard que celle-ci soit si peu présente dans les débats qui se déroulent actuellement dans le cadre de la campagne présidentielle. Ce débat a également le mérite de mettre en lumière les professions paramédicales, qui sont des acteurs essentiels de notre système de santé, notamment par rapport à cette problématique,

Toutes spécialités confondues, quatre-vingt-six départements enregistrent une baisse de la densité médicale sur la période 2007-2016. Le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous chez un médecin n'a cessé d'augmenter depuis cinq ; aujourd'hui, deux Français sur trois renoncent à des soins à cause des délais d'attente, contre 59 % en 2012. L'accès aux soins est à l'heure actuelle une préoccupation majeure de nos concitoyens, notamment dans les territoires ruraux. Toutes les analyses, toutes les études montrent que, avec le numérique, c'est la priorité principale de ces territoires. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable s'est penchée sur cette question

Dans ce document, nous avions souligné, parmi nos seize propositions, la nécessité de favoriser la coopération et la délégation entre les différentes professions de santé, de manière à alléger la tâche des médecins. Ce transfert de tâches permettrait de dégager du temps médical, afin que les médecins puissent se recentrer sur ce qui constitue le coeur de leur métier, le coeur de leur compétence. Ainsi, les infirmiers pourraient se voir confier l'accomplissement de certains actes, tels que les vaccinations. Les pharmaciens pourraient, de leur côté, contribuer au suivi des patients atteints de maladies chroniques.

Pour mettre en oeuvre ces transferts, il faut sortir d'une définition des professions de santé qui est établie sur des décrets de compétences rigides, en refondant les textes sur la base de la notion de missions, comme c'est déjà le cas dans un certain nombre de pays. Les progrès technologiques en matière de santé devraient également faciliter l'émergence de nouveaux partages de compétences entre les professionnels de santé. Le rôle des professions paramédicales est aussi essentiel

Je veux également attirer votre attention sur le fait que la plupart des professions de santé sont aujourd'hui l'objet d'une régulation en matière d'installation. C'est vrai depuis longtemps des pharmaciens, des kinésithérapeutes, des sages-femmes, des orthophonistes. Je rappelle que ce dispositif a permis d'augmenter de 30 % le nombre de kinésithérapeutes dans les zones sous-dotées entre 2012 et 2013. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, un certain nombre de mes collègues et moi-même proposons d'étendre le conventionnement sélectif aux médecins, en fonction de la nature des zones d'installation. Selon ce mécanisme, un médecin, pour s'installer dans une zone surdotée, devrait soit remplacer un confrère déménageant sur un autre territoire ou partant à la retraite, soit renoncer au conventionnement. Il s'agit non pas de coercition, mais de régulation d'une liberté, une liberté qui doit être soumise à un principe encore plus important : l'intérêt général. Les professions paramédicales ont montré la voie en matière de régulation d'installation. J'espère que nous saurons nous en inspirer pour faire face à la pénurie de médecins qui pose aujourd'hui de réels problèmes en termes d'accès aux soins et, au-delà, en termes d'égalité des territoires et de nos concitoyens. La parole La parole est à Mme Delphine Bataille, pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, chers collègues, ce débat soulève, une fois encore, la question essentielle des déserts médicaux qui concerne nombre de nos concitoyens des territoires ruraux qui l'accès aux soins de proximité reste difficile. Il nous invite également à réfléchir sur certaines solutions permettant de remédier à cette situation, tel le recours aux professions paramédicales. Les déserts médicaux sont des zones géographiques sous-dotées en professionnels ou établissements de santé ; cette pénurie touche de plus en plus de territoires et s'étend à toutes les spécialités médicales. Les zones rurales et hyper-rurales sont essentiellement concernées, mais les zones périurbaines, les petits bourgs éloignés des grands centres et certaines banlieues de grandes villes le sont aussi. Ce phénomène doit plutôt s'évaluer à l'échelle d'un bassin de vie. Il touche en particulier les territoires où vivent les populations les plus fragiles, qui souffrent d'une désertification économique et du désengagement des services publics. On peut ainsi trouver des déserts médicaux dans des départements- tel le Nord -qui s'inscrivent pourtant dans la moyenne nationale en matière d'accès à la santé. Dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, dont la densité médicale reste faible, ce sont, là encore, les territoires ruraux qui rencontrent de graves difficultés d'accès aux soins. Cette question est pourtant cruciale pour l'une des régions les plus peuplées de France et dont les indicateurs de santé, les plus bas à l'échelon national, demeurent inquiétants. Cela dit, dans la lutte contre la désertification médicale, madame la secrétaire d'État, il convient de saluer l'engagement du Gouvernement qui s'est traduit, dès 2012, par la mise en oeuvre du pacte territoire-santé, et qui a, par la suite, conforté et amplifié les résultats obtenus par un deuxième pacte en 2015. La loi de modernisation de notre système de santé a donné par ailleurs une assise législative à ces contrats territoriaux. La principale mesure- cela a été rappelé de nombreuses fois -concerne le développement des maisons et centres de santé pluriprofessionnels, dont le nombre a ainsi été multiplié par cinq depuis 2012, ce qui contribue à une réponse cohérente pour les professionnels de santé, bien sûr, mais aussi pour les usagers et pour les territoires fragiles. Les études les plus récentes montrent que les trois quarts des maisons de santé permettent de rééquilibrer l'offre de soins dans ces territoires. Cependant, ces équipements restent encore bien trop coûteux pour la plupart des collectivités locales. Les autres mesures principalement incitatives permettent d'encourager les médecins à s'installer dans les territoires sous-dotés, notamment le développement de formations plus adaptées et le soutien financier à l'installation dans les zones désertées. Si ces mesures se développent, elles sont coûteuses et nécessiteront beaucoup de temps pour résorber l'énorme déficit existant. De plus, de nombreux élus locaux sont aujourd'hui très inquiets, car leurs territoires, confrontés au vieillissement de la population, perdent de nombreux médecins, tendance à la baisse qui risque de s'accentuer dans les prochaines années. En effet, plus d'un médecin sur quatre a plus de 60 ans. Ce creux démographique est lié, bien entendu, au départ à la retraite de la génération du. Les élus doivent souvent faire face aux difficultés

des améliorations, mais il n'est toutefois pas évident que ces nouveaux futurs médecins se dirigent naturellement vers les territoires qui en ont le plus besoin. Ils privilégient avant tout leur vie familiale et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, refusant d'accomplir d'aussi longues journées que leurs aînés. Et les femmes, qui représentent dorénavant plus de 60 % des jeunes diplômés, préfèrent des horaires fixes et l'accès à un certain nombre de services de proximité. Sur ce point, il est évident que les territoires ruraux souffrent d'un manque d'attractivité par rapport aux villes. C'est pourquoi d'autres solutions sont souvent proposées, telles que le développement de la télémédecine qui ouvre la voie aux consultations, à la prise en charge et au prédiagnostic à distance. La mise en place de cette pratique n'est pas encore très développée, malgré le lancement d'un programme d'expérimentations prévu pour quatre ans sur neuf territoires pilotes. L'accès à la télémédecine pour les patients chroniques et pour les soins urgents est aussi un engagement du second pacte territoire-santé. De plus, la loi a conforté ce soutien à la télémédecine en prévoyant des dispositions destinées à clarifier son exercice, comme le partage d'informations entre professionnels. En clair, la télémédecine ouvre des perspectives intéressantes pour l'avenir, mais, là encore, cela prendra beaucoup de temps. Par ailleurs, le transfert de certaines activités médicales vers les professionnels paramédicaux constitue l'une des solutions majeures, tout le monde l'a bien dit. Cette idée n'est pas nouvelle elle est déjà mise en pratique dans d'autres pays. Les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, par exemple, ont pu organiser le transfert de certaines missions médicales à des infirmières praticiennes. En revanche, ce transfert est sûrement moins facile à mettre en oeuvre en France, car les médecins peuvent considérer que la qualité des soins risque de baisser, ou encore parce que les patients manifestent un manque de confiance à cet égard. Malgré les difficultés, le Gouvernement s'est engagé dans cette voie, permettant l'augmentation des missions pratiquées par les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les podologues, les opticiens, les sages-femmes, ainsi que la création d'un exercice en pratique avancée des auxiliaires médicaux. Tous ces postes sont exigeants et les candidats à ces formations sont recrutés sur des critères toujours très sélectifs. Pour aller plus loin, il faudrait peut-être non pas revoir globalement l'organisation de notre système, mais repenser certaines secteur paramédical. En conclusion, votre détermination, madame la secrétaire d'État, à endiguer le phénomène des déserts médicaux ne fait aucun doute, mais la plupart des mesures ne pourront résoudre à elles seules, en l'état actuel, le problème qui est bien plus étendu. Il convient notamment de privilégier, au-delà de la coopération interprofessionnelle que d'aucuns ont soulignée, une réflexion interprofessionnelle avec le ministère sur la démographie des acteurs de la santé.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, chacun sait que le phénomène des déserts médicaux s'intensifie dans bon nombre de territoires ruraux et de montagne en France et s'étend également au sein des agglomérations. De plus, dans son étude récente, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques souligne que, parmi les 62 000 médecins généralistes qui exercent en libéral, 15 000 environ ont plus de 60 ans et partiront à la retraite d'ici à cinq Dans le même temps, environ 10 000 médecins généralistes libéraux devraient s'installer. Plusieurs mesures incitatives tendant à favoriser l'installation des jeunes médecins dans les zones sous-dotées ont été prises, mais elles n'ont manifestement pas assez porté leurs fruits Considérant que la raréfaction des médecins est devenue inéluctable, il nous faut améliorer ou imaginer des alternatives. Aussi, face à cette problématique, nous pouvons nous féliciter de la tenue de ce débat, sur l'initiative de nos collègues de l'UDI-UC Quel rôle les professions paramédicales peuvent-elles jouer dans la lutte contre les déserts médicaux ? » En France, la profession paramédicale concerne une vingtaine de métiers, dont les infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, opticiens, orthophonistes, ambulanciers ... Il s'agit pour l'essentiel de professions de santé qui ne sont pas exercées par un médecin, une sage-femme, un dentiste ou un pharmacien. Une première piste consisterait à confier certaines tâches exercées par le médecin, voire certains actes, à d'autres professionnels de santé, telle la vaccination. On constate On constate souvent que les zones peu dotées en médecins généralistes sont également peu pourvues en spécialistes. De la même manière, on pourrait alors confier, par exemple, les renouvellements d'ordonnances des ophtalmologues aux opticiens.

Décloisonner les professions, sortir de la logique des décrets d'actes, optimiser les compétences des professions de santé et adapter les nomenclatures tarifaires, voilà autant de réformes de bon sens à mettre en oeuvre. Cela revaloriserait aussi le rôle des généralistes, qui pourraient alors se recentrer sur leur coeur de métier. Une deuxième piste est bien sûr de favoriser et faciliter l'exercice professionnel groupé dans des maisons de santé pluridisciplinaires ou pluriprofessionnelles. Ces maisons, regroupant plusieurs professionnels de santé sur un même lieu, vont dans le sens d'une coopération entre les professions médicales et paramédicales. Elles permettent une mutualisation des moyens, dont le local, le personnel administratif, mais aussi des compétences. Pour toutes ces raisons, les maisons de santé pluriprofessionnelles ont l'avantage de rassurer les jeunes médecins lors de leur installation.

permettent d'aller dans le sens d'un maintien de l'offre de soins dans les territoires sous-dotés en médecins. Aussi, on peut espérer que les ARS soient particulièrement attentives aux territoires dans la définition ou la mise à jour de leur schéma régional d'offre de soins puisque celui-ci établit les zones considérées comme fragiles en matière de démographie médicale et ouvre un droit aux projets de maisons de santé pluriprofessionnelles. Enfin, comment ne pas évoquer la télémédecine dans les domaines que sont la consultation, l'expertise, la surveillance et l'assistance, en y associant les professions médicales et paramédicales ? La télémédecine suppose néanmoins un effort de l'État et des opérateurs pour une couverture optimale du haut débit et de la téléphonie dans tous les territoires. La parole est à M.

plus que jamais indispensable d'exploiter tous les potentiels présents sur nos territoires et de reconnaître leurs intérêts. Afin de pouvoir assurer une offre de soins de qualité et de proximité, il nous faut absolument rattraper le retard existant en matière de maintien à domicile et de soins ambulatoires et reconnaître les professionnels du secteur paramédical comme maillon indispensable dans la prise en charge pluridisciplinaire des patients.

Les prises en charge à domicile, grâce à la coordination et à la transversalité entre établissements de soins et équipes de professionnels libéraux sur le terrain, sont maintenant mieux assurées. On voit enfin se développer une politique de maintien à domicile qui doit être une source d'économies sensible pour les prochaines années.

Ils apportent une réponse concrète aux attentes des patients et permettent une réorganisation des services de soins. Le développement de toutes les formes de coopération entre les professions médicales et paramédicales est indispensable si l'on souhaite élargir cette offre.

Nous ne sommes plus, dans ce pays, égaux par rapport à une offre de soins de proximité et de qualité. Il n'y a plus de gardes médicales le week-end et les jours fériés, les délais de rendez-vous sont souvent ahurissants.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le débat qui nous réunit ce soir nous propose de mettre en valeur les professions paramédicales et leur rôle dans les déserts médicaux. Je remercie le groupe de l'UDI-UC d'avoir

L'infirmière, l'aide-soignante et le kinésithérapeute sont indispensables, au côté du médecin, si l'on ne veut pas parler de désert médical. Les autres professions citées sont très utiles, mais il est possible de se rendre à leur cabinet, même s'il est éloigné,

Elle joue un rôle d'alerte, d'accompagnement, d'évaluation de la douleur, de soutien psychologique aux malades, aux aidants et à la famille. Elle effectue un certain nombre de soins fondamentaux

équilibre des anticoagulants, vérification des doses d'insuline des diabétiques, surveillance de la tension artérielle, prise de médicaments, prise du pouls, saturation en oxygène dans le sang, etc. Elle doit pouvoir joindre le médecin pour recevoir des conseils sur ces tâches qui lui ont été déléguées. L'infirmière et le médecin constituent un binôme parfaitement complémentaire, indispensable pour le malade.

encore que celle de l'infirmière. Le SSIAD est pour moi le socle de base fondamental du maintien à domicile ; les observations recueillies remontent à l'infirmière coordinatrice, qui peut les transmettre au médecin Le kinésithérapeute, quant à lui, joue également un rôle capital pour le maintien de la mobilité et de l'autonomie, la prévention des chutes et la rééducation respiratoire. Il observe la dégradation de l'état général, évalue la douleur et alerte le médecin en cas de besoin. Son rôle est essentiel dans les

États-Unis, Canada, Australie -ont fait apparaître des infirmiers praticiens qui proposent des consultations de première ligne et des prises en charge de problèmes mineurs, et qui orientent le patient au sein du système de santé ou pour le suivi des maladies chroniques. Certains universitaires, en France, ont évoqué la possibilité pour les infirmiers, au terme d'une formation complémentaire, de remplacer le médecin le médecin pour le renouvellement d'ordonnance, lorsque le malade est stabilisé et qu'il n'a pas de nouvelles pathologies. À titre personnel, j'y suis absolument défavorable, car une consultation ne doit pas se traduire simplement par une signature au bas d'une page de renouvellement. La consultation est un lieu d'échanges entre le médecin et le patient

les jeunes praticiens médicaux et paramédicaux souhaitent travailler ensemble, se parler, se rencontrer pour optimiser leurs relations de travail. L'implantation de maisons de santé pluridisciplinaires, avec un projet de soins et de santé, constitue une incitation forte pour l'installation

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la lutte contre les déserts médicaux est un sujet qui me préoccupe. La Mayenne est le troisième plus important désert médical de France.

concerne la mise en place d'un observatoire, l'animation de travaux d'enquête auprès des professionnels, la mise en lien de tous les acteurs a été fédérateur et a permis une vision départementale.

Dans la plupart des territoires, ces derniers se sont entourés de tous les acteurs institutionnels du champ sanitaire et médico-social, ainsi que des associations d'usagers. La création de maisons de santé pluridisciplinaires a également pu s'orienter sur des pôles de santé adossés à un hôpital local, voire à des EHPAD. Le partage de pratiques et de ressources entre professionnels de santé est alors une culture d'exercice qui permet une meilleure coordination entre personnel médical et paramédical. Il facilite les coopérations et intègre la médecine de ville dans les organisations de soins sur le territoire.

La notion de parcours a, dans de tels dispositifs, tout son sens et prend appui sur le contrat local de santé qui détermine les besoins spécifiques du territoire. C'est, par exemple, la présence d'un médecin spécialiste du diabète qui assure des permanences au sein d'un pôle santé et qui s'appuie le reste du temps sur les médecins et les infirmières travaillant sur le site. C'est aussi l'appui d'un spécialiste par télémédecine pour un diagnostic plus avancé en chirurgie reconstructrice, qui s'appuie ensuite sur le travail d'un masseur-kinésithérapeute. C'est encore la plus-value apportée par les contrats souples passés avec de jeunes médecins, sous le statut d'assistant libéral, qui leur permettent d'appréhender en douceur l'exercice libéral. C'est enfin le cas des professionnels de la protection maternelle et infantile, sages-femmes et puéricultrices, qui viennent s'ajouter à l'effectif d'une maison pluridisciplinaire. Tous ces exemples parmi d'autres mettent en exergue le décloisonnement nécessaire à cette nouvelle approche professionnelle. Il convient également de faciliter l'exercice professionnel. À cet égard, la mise en place de maisons de santé ou de pôles de santé a permis aussi de réfléchir à l'accueil des patients et à leur suivi administratif. L'embauche de personnel dédié et mutualisé répond pleinement à cette question et décharge les médecins, notamment, de tout ce temps consacré aux charges administratives. De plus, il a été mis en place en Mayenne, depuis 2006, un accueil coordonné pour l'inscription des médecins au tableau départemental, répondant ainsi à l'attente des praticiens et visant à simplifier réellement les démarches administratives. En conclusion, et par expérience, je témoigne donc que les professions paramédicales ont un rôle essentiel dans la lutte contre les déserts médicaux. Mais il faut les associer pleinement à la réflexion pour trouver une réponse d'accès aux soins coconstruite sur les territoires. Néanmoins, pour lutter contre la désertification médicale, cela ne suffit pas, bien évidemment

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la santé constitue aujourd'hui l'une des premières préoccupations des Français. Ainsi, dans les Pays de la Loire, lors de l'élaboration du pacte « ruralité » de juin 2016, ce fut, avec l'accès au numérique, la deuxième préoccupation citée.

Face à des besoins croissants- forte natalité, vieillissement accéléré de la population -, on a constaté une double fracture sanitaire, avec une tension tant sur les effectifs que sur les conditions d'exercice des professionnels de santé de proximité, ce dans les zones rurales, périurbaines et même dans certains quartiers de ville. De plus, l'exercice des professionnels de santé dans les territoires est modifié, avec la recherche d'un meilleur équilibre entre vie familiale et vie professionnelle, la volonté de travailler en réseau, les évolutions technologiques- télémédecine, médecine prédictive et personnalisée le passage d'un système de santé centré sur la logique curative à un système plus soucieux de prévention. La révolution numérique en cours va évidemment renforcer un exercice pluriprofessionnel au service d'un patient davantage responsabilisé. L'enjeu principal pour les élus est d'encourager le maintien et l'installation durable des professionnels de santé dans les territoires qui en manquent aujourd'hui ou qui en manqueront demain, en coordination avec les nombreux acteurs déjà fortement mobilisés. La loi HPST avait déjà institué une approche globale de la prise en charge du patient. Le rôle du médecin généraliste est donc renforcé en tant qu'acteur pivot de première ligne. Mais il convient de ne pas se focaliser uniquement sur les généralistes, dans la mesure où leur travail est en forte interaction avec les autres avec les autres professions de santé- infirmiers, kinésithérapeutes, pharmaciens, sages-femmes, etc. -et le secteur médico-social. La démographie est très variable selon la profession concernée. En Pays de la Loire, les sages-femmes formées seraient très, voire trop nombreuses À cet égard, notre plan régional s'appuie, entre autres, sur plusieurs leviers. Il s'agit, tout d'abord, de stimuler les innovations, celles qui touchent l'organisation des modes d'exercice des professionnels de santé comme les innovations numériques et technologiques permettant de contribuer à mettre la santé digitale au service des patients. des patients. Les maisons de santé pluriprofessionnelles constituent ensuite une réponse à l'évolution des modes d'exercice souhaitée. Mais sans diagnostic ni organisation préalable des élus et des professionnels autour des priorités de santé d'un territoire, initiatives et investissements sont voués à l'échec, comme en témoignent certaines maisons de santé pluriprofessionnelles devenues des coquilles vides. Cela demande du temps, de l'énergie et de la méthodologie qui font parfois défaut sur certains territoires, notamment fragilisés. Par ailleurs, le maintien d'une dynamique pluriprofessionnelle n'est jamais acquis, ce qui requiert aussi un soutien à certaines démarches déjà engagées nécessitant d'être confortées ou redynamisées.

Nous envisageons aussi, dans les lycées et centres d'apprentissage, des interventions d'étudiants en médecine ou en formation paramédicale, en partenariat avec l'ONISEP. Le quatrième levier repose sur la formation. Un bon maillage des instituts de formation sanitaire et sociale permet aux jeunes et aux et aux adultes intéressés par ces métiers, mais confrontés à des problèmes de mobilité, de pouvoir s'engager dans ces formations qui peinent de plus en plus à recruter. Il permet aussi aux employeurs locaux de pouvoir tisser des relations avec ces instituts et de faciliter ainsi l'accueil en stage puis le recrutement. Les futurs soignants doivent être sensibilisés dès leur formation à l'exercice pluriprofessionnel : partage de locaux entre filières de formation différentes, cours en commun, partage de formateurs et de lieux de stage, événements organisés en commun ... À titre d'exemple, je citerai la mutualisation des moyens et des ressources, y compris des locaux, sur l'agglomération du Mans,

La région conditionne aussi son soutien aux maisons de santé à l'accueil de stagiaires étudiants en médecine ou en instituts de formation sanitaire. La prise en compte du vieillissement Les territoires dont l'offre de santé et de proximité est la plus fragilisée sont bien souvent ceux qui comptent une population vieillissante plus importante que la moyenne, entraînant des besoins de soins et de prévention croissants.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la désertification médicale touche l'ensemble de notre pays, et bien sûr mon département, les Côtes-d'Armor. Les déserts médicaux ne sont plus seulement des zones déficitaires en services, haut débit ou commerces. La ville de Lamballe, où passe le TGV, perd successivement ses généralistes, qui ne sont pas remplacés.

Je veux rendre hommage à Hervé Maurey, qui mène sur le sujet un combat déterminé au sein de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Je le soutiens totalement. Non, les solutions purement incitatives proposées depuis des années ne sont pas suffisamment efficaces. Il nous faut, après avoir perdu tant de temps en tergiversations, prendre de réelles mesures, qui auront pour objectif de résoudre ces difficultés à court, moyen et long terme. Madame la secrétaire d'État, les solutions que nous devons apporter relèvent non pas simplement des syndicats et ordres professionnels, mais aussi du législateur et des élus locaux dans le cadre de l'aménagement du territoire. Certes, cela doit se faire en concertation, mais avec courage et détermination. Récemment, mais bien tardivement, dans la perspective de l'élection présidentielle, le conseil de l'Ordre a fait dix propositions, développées hier- est-ce un hasard ? -à l'occasion d'un débat dans ses locaux. La régionalisation du me paraît une bonne idée. Cette idée de partir des territoires est d'ailleurs l'une des conclusions du groupe de travail de l'AMF22, Cela permettrait de conserver les jeunes médecins dans le périmètre de leur lieu d'études, là où ils auraient fait leur stage. Actuellement, en Bretagne, le nombre de médecins formés chaque année couvre à peine les besoins en la matière des collectivités, hôpitaux, cliniques et établissements publics divers. Les lobbies sont Les lobbies sont puissants. Nul n'a jamais touché au principe de la libre installation. Dernièrement, à l'Assemblée nationale, la commission des affaires sociales avait adopté un amendement, finalement rejeté en séance avec un avis défavorable de la ministre Marisol Touraine, qui fut pourtant cosignataire, lorsqu'elle était dans l'opposition avant 2012,

les élus ont soutenu vivement le premier vice-président du conseil départemental, qui demandait avec force et vigueur que soit remise en cause la liberté d'installation. Ce n'est pas ce que je propose. En revanche, il n'est plus acceptable que profession, Ordre et syndicats n'acceptent pas que nous arrêtions d'autoriser de nouvelles installations de médecins conventionnés dans les secteurs géographiques de notre pays qui sont surdotés. qui sont surdotés. Ceux-ci devraient être délimités, bien entendu en étroite collaboration avec la profession, et réactualisés chaque année. Il y a, bien sûr, les maisons de santé pluridisciplinaires, mais elles ont un coût, supporté par les collectivités.

bien entendu en étroite collaboration avec les professionnels. Il faut aussi que les professions paramédicales puissent se voir reconnaître le droit de pratiquer tout acte qui ne nécessiterait pas l'intervention et la compétence d'un médecin. L'article 119 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 prévoit ainsi l'extension des compétences des professions paramédicales. Mais il faut un décret d'application, dont la parution est aujourd'hui très attendue. Il serait, paraît-il, reporté en 2018 ... Pourquoi ? J'évoquerai en particulier le rôle des infirmiers et infirmières, qui sont soumis depuis 2008 à des règles contraignantes d'installation sur le territoire permettant une couverture homogène. et des infirmières cliniciens en formation initiale ou continue pour les professionnels en activité permettrait d'assurer des tâches aujourd'hui dévolues aux médecins, lesquels se concentreraient sur les actes essentiels de la médecine. Des pays anglo-saxons et scandinaves ont poussé plus loin la logique de coopération. Le bilan des dispositifs en question en termes d'accès aux soins et de prévention est très positif, pour la plus grande satisfaction des usagers.

notamment pour le patient. Mais ne pourrait-on pas envisager que le médecin coordonnateur, en lien avec le médecin généraliste, puisse faire des renouvellements d'ordonnance dès lors qu'il n'y a pas lieu de changer la prescription, d'y ajouter ou d'en retirer des médicaments ? Il y a Il y a des mesures simples et concrètes à prendre immédiatement ! C'est une question de bon sens et de volonté. Je veux enfin insister sur la nécessité de laisser une certaine souplesse d'organisation aux acteurs sur le terrain, en évitant tout dogmatisme ou tout corporatisme qui, pour le moment, contribue à empêcher d'apporter des solutions rapides à la désertification médicale. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le constat est connu depuis longtemps et devient véritablement alarmant : l'accès à un médecin généraliste ou spécialiste est, sur certains territoires, de plus en plus difficile. Cela résulte de deux phénomènes : d'une part, les départs à la retraite de nombreux professionnels de la génération du baby-boom sans que l'assouplissement du ait encore pleinement produit ses effets-

plus, l'allongement de la durée de la vie et le vieillissement de la population vont conduire à des besoins croissants. C'est pourquoi je suis convaincu que, au-delà des mesures « rustines », ou plutôt « pansements », en l'occurrence, il est indispensable de repenser l'ensemble de la chaîne de santé et les missions des différentes professions médicales et paramédicales. Il s'agit non pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul, mais plutôt de tirer tout le monde vers le haut-

Dès lors que le médecin continue de superviser les soins et qu'il est rémunéré pour cela, il n'est en rien infamant, pour aucun des acteurs, que certaines missions puissent être réalisées par des professionnels paramédicaux, d'autant que le développement des regroupements et de la coordination rend possibles ces évolutions. Sinon, faute d'ophtalmologistes, faut-il se résoudre à des délais de plusieurs mois ? En la matière, on voit bien que la clé est plutôt à chercher dans une meilleure articulation avec les orthoptistes.

l'avenir est à la prévention ; les professions paramédicales y joueront certainement un rôle majeur. Certains de nos voisins sont allés très loin dans le transfert de certaines activités médicales. Je pense à la Grande-Bretagne, où les infirmières interviennent dans le dépistage, les bilans de santé ou le suivi des malades chroniques.

Tout au long du quinquennat, nous avons eu l'occasion de débattre, dans cet hémicycle, de cette question centrale, qui- reconnaissons-le ! -dépasse largement les clivages partisans habituels.

Ils sont aussi inquiets face au parcours du combattant qu'il faut parfois accomplir pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste. Ces enjeux sont devenus une préoccupation majeure pour nos concitoyens et une priorité pour le Gouvernement. pourquoi, au nom du Gouvernement, je veux remercier le groupe de l'UDI-UC d'avoir inscrit ce débat à l'ordre du jour de votre assemblée et d'avoir choisi de mettre en avant un aspect concret, concret, pragmatique, dans la réponse à apporter pour lutter contre les déserts médicaux : la place et le rôle qu'ont à jouer les professions paramédicales. Notre système de santé

Nous le savons tous, la problématique de l'accès aux soins va bien au-delà de la question des consultations médicales. Aujourd'hui, le vieillissement de la population, le développement des maladies chroniques, la complexité des prises en charge nous imposent de faire évoluer notre vision de l'accès aux soins.

y compris lorsque le patient est en situation dite complexe ou de handicap ou qu'il se trouve en perte d'autonomie. C'est pour répondre à cet enjeu que le Gouvernement agit depuis 2012. Réduire les inégalités territoriales de santé a été l'une des grandes priorités de l'action de la ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine. Nous avons agi non seulement pour mieux répartir l'ensemble des professionnels, mais aussi pour réorganiser le système de soins. D'abord, nous avons renforcé le travail d'équipe : dès la formation, nous avons développé cette culture. Vous le savez, les professions de santé s'apprennent sur les lieux du futur exercice. Un enseignement exclusivement hospitalier est un frein à la naissance de vocations pour l'exercice en ambulatoire, encore plus dans les déserts médicaux. Absolument ! C'est pourquoi la loi de modernisation de notre système de santé a permis d'élargir les lieux pouvant être agréés comme terrains de stage. Désormais, un infirmier, un pédicure-podologue ou un kinésithérapeute peut réaliser une partie de sa formation dans des maisons de santé pluriprofessionnelles, des centres de santé ou des cabinets de professionnels libéraux. Pour mieux accompagner au quotidien chaque professionnel de santé, qu'il soit médical ou paramédical, je vous rappelle aussi qu'un portail d'accompagnement des professionnels de santé a été ouvert dans chaque région, afin d'apporter aux jeunes et aux professionnels toutes les informations pratiques sur la formation, l'installation et les aides proposées, ainsi que sur les conditions d'exercice. Je veux ensuite, évidemment, évoquer les maisons de santé pluriprofessionnelles. L'étude de recherche et documentation en économie de la santé, conduite en 2014, a clairement montré que l'implantation des maisons de santé permettait de maintenir et même de développer l'offre de soins dans les territoires à dominante rurale, plus fragiles. Ces structures regroupées, qui associent des professions médicales et paramédicales autour d'un même projet de santé, dans un même lieu, ont fait la preuve de leur attractivité. Nous voyons bien qu'elles correspondent fortement aux attentes des patients, en regroupant tous les professionnels sur un seul site et en garantissant ainsi une meilleure continuité des soins.

Deuxième chantier d'importance, celui de la définition de parcours de soins, dans lesquels les professions paramédicales ont une place centrale. L'une des ambitions de la loi de modernisation de notre système de santé est de faciliter au quotidien les parcours de santé des patients, en organisant un premier recours efficace. Ainsi, la mise en place d'équipes de soins primaires et des communautés professionnelles territoriales de santé doit permettre de faciliter les parcours de soins dans les zones à faible densité grâce à la coordination des professionnels de santé. Concrètement, les communautés les maisons de santé, les professionnels de santé de premier et second recours, les travailleurs sociaux et les professionnels médico-sociaux, afin d'assurer une meilleure coordination de leur action respective, de structurer des parcours de santé et d'améliorer la couverture des territoires par des équipes de soins primaires.

coordination autour d'un patient âgé n'est possible dans de bonnes conditions que si l'organisation des professions de santé sur un même territoire a été adaptée pour anticiper les situations de rupture.

Ce dispositif s'adresse aux personnes âgées de 75 ans et plus, dont l'autonomie est susceptible de se dégrader pour des raisons d'ordre médical ou social. Afin de préserver l'autonomie des personnes âgées, la démarche engagée dans le cadre du programme PAERPA renforce notamment la prise en charge à domicile, en s'appuyant sur tous les professionnels de soins primaires médecins traitants, infirmiers, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes et autres auxiliaires médicaux. Si la coordination des professionnels de santé est un facteur essentiel d'une bonne prise en charge des patients sur l'ensemble du territoire et permet un parcours de soins plus lisible,

Ce dispositif est d'ores et déjà une réussite. Au mois de novembre 2015, 300 000 patients avaient bénéficié d'un suivi et d'éducation thérapeutique dans son cadre. À la fin de l'année 2016, 1 441 médecins travaillaient en collaboration avec l'un des 416 infirmières

Cette actualisation, attendue par les professionnels, constituera une étape très importante. Les discussions, qui ont commencé au début du mois de février, porteront notamment sur la possibilité d'étendre les compétences des infirmiers en matière de vaccination.

Les orthoptistes constituent les principaux acteurs de cette démarche, en coopération avec les ophtalmologues. Un contrat collectif, proposé aux structures de soins coordonnées- centres et maisons de santé permettra d'apporter un soutien financier pour investir dans du matériel, afin de permettre des consultations d'orthoptie réalisées sur délégation d'un ophtalmologiste. Cela permettra par exemple à l'orthoptiste d'effectuer le dépistage de la rétinopathie diabétique comme un bilan visuel.

pour inciter à exercer dans un établissement d'un territoire présentant un risque de fragilisation de l'offre de soins, c'est-à-dire dans les zones sous-dotées. Cette mesure devrait d'abord concerner les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes.

leur pratique quotidienne. Au-delà de la théorie, ces professionnels sont demandeurs de solutions concrètes, palpables. C'est le sens du travail que nous avons engagé durant les cinq dernières années. Nous n'avons pas la prétention d'affirmer que